L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle

dédiées au portage foncier, dans le souci d'une plus grande transparence du marché foncier. Simplement, nous avons souhaité élargir la liste des exceptions à cette nouvelle règle. Ainsi, un amendement avait été adopté

afin de favoriser l'installation en agriculture ou de permettre la préservation des exploitations agricoles existantes sur notre territoire. Nous avons aussi conservé la disposition permettant aux SAFER de détenir plus de 30 % des parts d'un groupement foncier agricole ou d'un groupement foncier rural, ainsi que la disposition les autorisant à maintenir leur participation au capital d'une société durant un maximum de cinq ans, comme cela existe pour la détention de terres, afin de leur permettre de mieux exercer leurs missions de portage du foncier, lorsque ce portage s'effectue par le truchement de l'acquisition de parts d'une personne morale. De la même manière, nous avons maintenu la disposition obligeant à conserver cinq ans les parts sociales attribuées en contrepartie d'apports en terres à une société, afin d'éviter le contournement des règles sur le foncier agricole. Les articles 6 et 7, qui concernent respectivement le barème de la valeur vénale des terres et l'assouplissement des concessions temporaires d'utilisation de terres agricoles en l'attente d'aménagements par les collectivités territoriales, ont été adoptés sans modification.

que nous avions votée, faute de consensus sur ce point dans le milieu agricole, mais surtout afin d'éviter de casser ce qui marche encore dans 50 % des départements. La CMP a aussi restreint le champ de la nouvelle exception que nous avions introduite à l'obligation de passer par une société de portage foncier pour les acquisitions de terres par les personnes morales. Les députés craignaient une perte de substance de la nouvelle obligation de passer par une filiale pour des acquisitions de terres : des sociétés auraient pu louer des terres à seule fin de pouvoir en faire l'acquisition directement ensuite. Une rédaction de compromis a permis de n'exonérer de l'obligation de passer par une société de portage foncier que pour les acquisitions de terres agricoles louées par des sociétés en vertu d'un bail conclu avant 2016.

Ainsi, nous prenons toutes les précautions pour empêcher le contournement de la règle dans le futur. Un débat subsistait sur la date de mise en application des nouvelles règles

Au final, nous nous sommes entendus sur une application des nouvelles règles d'un seul bloc, c'est-à-dire de l'ensemble des articles de cette loi, trois mois après la promulgation de la loi. Le volet concernant les produits phytopharmaceutiques n'était pas consensuel non plus à l'issue des lectures à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. D'ailleurs, monsieur le ministre, vous aviez largement évoqué le sujet en première lecture. Vous étiez sur la pénalisation ; moi, j'étais sur l'encouragement sur l'encouragement ! Sur les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, les CEPP, nos approches étaient très divergentes. Le Sénat, considérant qu'il s'agit d'un dispositif expérimental, avait supprimé la disposition sur les sanctions financières encourues par les distributeurs en cas d'insuffisance de certificats accumulés au terme de l'expérimentation. Nous préférions des mécanismes d'incitation et d'encouragement plutôt que des sanctions. Le rapporteur de l'Assemblée nationale a insisté sur le fait que l'absence de sanctions dévitalisait un peu le dispositif et ne permettrait pas- au contraire ! -de récompenser les « bons élèves ». Nous avons Nous avons aussi pu constater que la sanction ne touchait pas directement les agriculteurs, et même que les agriculteurs, en lançant des actions en faveur de techniques alternatives aux produits phytopharmaceutiques classiques, pouvaient aussi engranger des CEPP et les valoriser en se les faisant racheter par les distributeurs.

En cas de pression parasitaire forte, nous avons l'assurance que le mécanisme mis en place ne pénalisera pas l'utilisation des produits nécessaires et dans les quantités nécessaires, même si elles sont importantes, pour éradiquer insectes, champignons ou encore plantes adventices.

En CMP, nous nous sommes donc mis d'accord pour réintroduire la sanction financière des distributeurs, mais après une évaluation complète de l'expérimentation des CEPP, qui aura lieu en 2020.

et dans les parcs et jardins des particuliers, le Sénat avait introduit avec l'article 8 A, une dérogation générale jugée un peu trop large par le rapporteur de l'Assemblée nationale et par vous, monsieur le ministre.

Sur cette proposition de loi, nous avons cherché à travailler dans un esprit constructif, pour trouver des solutions pragmatiques à de vrais problèmes, au-delà des clivages partisans. La question du foncier agricole reste cependant encore largement ouverte. Si nous voulons que les paysans restent maîtres de la terre indispensable à toute production,

C'est une tâche à laquelle je vais m'atteler, en lançant des consultations pour établir un état des lieux plus complet sur la détention et l'utilisation des terres agricoles, avant de proposer les solutions pérennes, dont notre agriculture a tant besoin, dans une future loi foncière. La définition du statut de

L'outil de la négociation, l'outil de la gouvernance des SAFER est un point d'équilibre très important pour assurer cet accès au foncier, limiter les risques d'inflation sur cet accès et, en même temps, résister

à ces certificats d'économie de produits phytosanitaires. Je vois d'ailleurs renaître souvent des débats sur les découplages entre conseil et vente, afin d'essayer de résoudre le problème. Les certificats d'économie de phytosanitaires sont la meilleure réponse.

à mettre sur la table des outils nouveaux qui permettront d'atteindre les objectifs de baisse des phytosanitaires sans faire payer quoi que ce soit aux agriculteurs. Ces méthodes et ces dispositifs nouveaux offrent une perspective à l'agriculture

de l'agroécologie, qui offre des perspectives environnementales et surtout économiques, mais aussi une vraie revalorisation du métier d'agriculteur. Les agriculteurs sont parties prenantes des grands enjeux de la société, à la fois, parce que ce sont des producteurs d'aliments-

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, aujourd'hui, je suis très satisfait, en tant que sénateur et en tant qu'agriculteur. Le consensus trouvé dans le cadre de la commission mixte paritaire prouve que, au-delà de nos différences, de nos convictions politiques, nous pouvons nous unir pour des objectifs communs : la préservation d'un modèle d'agriculture familiale et une réponse à l'attente sociétale s'agissant de la baisse des produits de traitement. Je tiens tout particulièrement à remercier les rapporteurs, MM. Gremillet et Potier, qui ont su établir un contexte d'échange serein et, surtout, constructif. Le succès de la CMP repose sur un double accord : un accord de raison et un accord de coeur. Je commence par l'accord de raison. Nous avions essentiellement trois points de divergence sur les articles 1, 8 et 10. Ils ont fait l'objet de débats, dans le seul intérêt général. Concernant le foncier et l'article 1 de cette proposition de loi, notre objectif commun est bien de diminuer la spéculation foncière et la dilapidation de terres à des investisseurs étrangers. Il n'est nullement dans notre intention de nous attaquer aux formes sociétaires en général. Jérémy Decercle, président national des Jeunes Agriculteurs, indiquait récemment que deux jeunes sur trois choisissent cette entité juridique lors de leur installation. La majorité de ces modèles sont vertueux et revêtent de nombreux avantages : mutualisation de moyens matériels et humains, transmission progressive de l'exploitation, protection du patrimoine personnel. La CMP a donc trouvé un accord sur les amendements sénatoriaux précisant le dispositif, sans pénaliser les exploitations existantes, quelles que soient les formes sociétaires. Le droit de préemption des terres agricoles est maintenu aux sociétés titulaires d'un bail conclu avant le 1 janvier 2016, sans obligation de création d'une société de portage. Non, il s'agissait uniquement de moraliser les transactions, en comblant un vide juridique et en repositionnant le rôle des SAFER. L'affaire des terres vendues dans l'Indre a permis un focus médiatique et une réaction des pouvoirs publics, mais il ne faut pas que cette actualité nous fasse oublier le problème majeur du foncier : l'artificialisation des terres pour des logements, des zones industrielles ou commerciales ou des routes. Les chiffres sont affolants et tournent en boucle sur le : près de 80 000 hectares disparaissent, en moyenne, chaque année, soit l'équivalent d'un département tous les sept ans ou une perte de trois exploitations par jour.

Autant de raisons qui poussent un exploitant à profiter de l'aubaine financière que peut représenter la vente de ses terres. Si les causes sont humaines et compréhensibles, les conséquences en sont énormes et diverses. D'abord, cette artificialisation induit la perte de sols fertiles, qui bénéficient quelquefois d'une irrigation financée par des deniers publics. Puis, elle met en péril notre indépendance alimentaire, l'Europe important l'équivalent de la production de 35 millions d'hectares. Ensuite, elle a un impact direct sur la biodiversité : les sols stabilisés deviennent imperméables, ce qui a des effets évidents sur le cycle de l'eau. on le constate régulièrement avec les phénomènes d'inondation que subissent nos différents territoires. Comment enrayer ce phénomène d'artificialisation ?

C'est crucial. Nous devons soutenir ces sociétés, notamment sur leur volume de ventes annuelles et sur la question du stock de foncier. Ces stocks leur sont indispensables pour effectuer un remembrement, qui est nécessaire aux installations et au renouvellement des générations. Les SAFER ont massivement déstocké pour équilibrer leur budget. Ainsi, dans l'ancienne région Languedoc-Roussillon, le marché du foncier agricole s'est effondré en 2007, avec la crise viticole

Si les outils juridiques et législatifs existent, nous devons nous intéresser à la volonté politique et au financement des portages. Je redis ma proposition de flécher une partie de la taxe spéciale d'équipement récoltée par les établissements publics fonciers vers les SAFER, par territoire et une convention d'objectifs. Je laisse cette proposition à la discussion et à l'étude. deuxième partie de la proposition de loi a créé un débat : les articles 8 et 10, qui concernent spécifiquement le développement du biocontrôle. Là encore, nous sommes parvenus à un consensus, car l'idée n'est pas de figer des activités de la filière. Il s'agit d'offrir aux agriculteurs, premiers touchés par les pesticides, et aux consommateurs une réponse raisonnée aux objectifs de santé publique et de protection de l'environnement. Nous avons décidé la mise en place d'expérimentations et d'évaluations. Elles permettront d'analyser l'efficience des mesures préconisées. La commission mixte paritaire a également intégré une exception à l'interdiction faite aux collectivités territoriales d'utiliser des produits phytopharmaceutiques classiques

le directeur a insisté sur la nécessaire pédagogie des agriculteurs pour mieux appréhender l'évolution des pratiques. Dans les faits, les vendeurs répondent souvent strictement aux demandes des professionnels. Et la réalité est parfois inquiétante : les appareils de traitement ne sont pas forcément bien réglés ; les produits sont parfois suremployés, avec des dosages qui ne correspondent pas toujours à la surface réelle exploitée.

Les vendeurs, qui bénéficient de trois années pleines pour faire évoluer leur offre de produits et développer les conseils, devront comprendre, avec raison, les enjeux tout aussi environnementaux que sociétaux. Cette activité de conseil ne doit pas déboucher sur une augmentation du coût des produits, que les exploitations ne pourront pas supporter. Si les agriculteurs sont affaiblis, cela atteindra à terme leur propre activité.

Ils ne supportent plus les clivages politiques et les querelles de clocher qui sclérosent les décisions. L'efficacité est un triptyque simple : un problème, une solution, une action ! Nous ajoutons l'évaluation, condition demandée par les chefs d'entreprise et les citoyens pour accepter les contraintes générées. Si nous produisons des lois dans un but d'amélioration, nous nous devons d'en étudier l'impact pour coller à la réalité. La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme nous l'avions souligné lors des débats en première lecture, la spéculation sur le foncier agricole et forestier n'est pas propre aux pays du sud. C'est une terrible réalité que connaissent aujourd'hui tous nos territoires. En effet, après la forêt et les grands vignobles, ce sont les terres intermédiaires qui sont aujourd'hui dans la ligne de mire d'investisseurs peu scrupuleux, ou trop gourmands.

le mouvement actuel provient de la dérive individualiste de la course à l'agrandissement, d'un relâchement du contrôle des structures, de brèches législatives ouvertes en 2006 et de l'arrivée de fonds spéculatifs à partir de 2008. C'est pourquoi nous nous réjouissons des travaux de la commission mixte paritaire. Nos deux assemblées ont réussi à trouver un accord satisfaisant

et le recours croissant à des entreprises de travaux agricoles, ce qui remet en cause le modèle d'agriculture familiale. La financiarisation des terres est bel et bien en marche- tout n'est pas nécessairement « en marche », mais ça, oui ! -, ce qui conduit à l'élimination des petits exploitants et met une très grande partie de la profession en difficulté. le nombre des fermes de moins de dix hectares a diminué de 56 % en une décennie, passant de 340 000 en 1990

Presque ! Or, nous le savons, la politique foncière est un pilier de toute politique agricole et alimentaire. Elle participe à l'orientation globale de notre modèle agricole et à la structure des exploitations sur le territoire national. Elle est aussi un enjeu important pour le renouvellement et l'installation de nos jeunes agriculteurs, trop souvent confrontés à des problèmes touchant au foncier, lorsqu'ils commencent leur activité professionnelle. C'est pourquoi il nous aurait semblé nécessaire que le Gouvernement soit porteur d'un grand projet de loi sur le foncier agricole, en lieu et place de mesures ponctuelles et éparses. Cela devra être un chantier législatif prioritaire, quel que soit le prochain Gouvernement. Comme cela a été dit lors des débats, pour le moment, on corrige des failles législatives introduites voilà une dizaine d'années. Mais contrer ce mouvement libéral de concentration des capitaux n'est pas à la hauteur des enjeux. Le foncier doit être redécouvert comme un élément commun, commun, régulé par la puissance publique. De nombreuses questions restent en suspens. Ouvrir le droit de préemption des SAFER sur les parts de société doit s'accompagner d'une redéfinition de leurs missions, comme l'intégration du contrôle des structures. Il Il faudra aussi s'attaquer à la redéfinition de leurs moyens d'action, de leur statut, avec une possible transformation en établissement public, et de leur financement, afin de leur éviter de rechercher des fonds propres. Nous devrons également

C'est d'ailleurs le sens de la proposition de loi de revalorisation des retraites agricoles de nos collègues du groupe GDR de l'Assemblée nationale, qui a été adoptée récemment. De même, il est indispensable d'encadrer De même, il est indispensable d'encadrer les prix des terres, de sorte qu'ils soient en corrélation avec le revenu agricole qui peut en être dégagé. Ne pas Ne pas le faire conduirait inéluctablement à de très grandes difficultés pour l'installation des jeunes. L'étalement urbain et la concentration sans précédent des terres cultivables aux mains de grosses exploitations participent à la disparition des paysans. Alors que l'opacité règne sur les transactions foncières, la logique financière se répand. Si nous ne faisons rien de plus, ce sont des qui contrôleront demain les campagnes françaises. Nous ne le voulons absolument pas Sur le second volet de ce texte, le biocontrôle, il y a des avancées positives. Mais, là encore, il faudra y revenir, car la procédure législative accélérée ne nous permet pas de faire un travail de fond

Je salue la sagesse des députés. Ils se sont ralliés à la rédaction du Sénat pour les articles 8 et 9, qui allègent les exigences pesant sur les professionnels utilisant des techniques alternatives. Le dernier désaccord portait sur la disposition la plus importante, l'article 10,

L'achat de terres agricoles par des investisseurs étrangers, notamment dans le département de l'Indre, a suscité une grande inquiétude parmi les acteurs du monde agricole et a contribué à sensibiliser l'opinion publique. Mais, à mon sens, cela ne suffit pas pour déclencher une nouvelle législation. Plus qu'un enjeu économique, le phénomène d'accaparement des surfaces agricoles représente aujourd'hui un enjeu d'avenir pour notre pays. Les terres agricoles représentent notre capacité à produire et à assurer notre souveraineté alimentaire, mais il est aussi question du travail et des revenus et des revenus de nos agriculteurs. L'agriculture est également un outil de rayonnement de la France sur la scène internationale. Elle est l'un des emblèmes de notre pays, auquel nous sommes tous profondément attachés. C'est pourquoi il est primordial de mener une politique capable de garantir l'émergence d'un modèle agricole français compétitif et durable. Au-delà de la question de la revente des terres agricoles que nous examinons dans cette proposition de loi, il est donc aussi important de revoir les questions de transmission des exploitations. Sur le fond, cette proposition de loi constitue un texte d'ajustement. Notre groupe l'accueille favorablement, puisqu'il essaie de répondre aux dysfonctionnements de la régulation de ce marché. Je ne reviendrai pas sur les différentes mesures. Ce texte permet de combler les lacunes juridiques existantes, qui ont contribué aux dysfonctionnements observés ces derniers mois. Cependant, nous regrettons que cette question n'ait pas fait l'objet d'un texte plus large relatif à la politique foncière. L'accumulation de petites réformes crée un manque de cohérence et de clarté. les discussions ont permis de corédiger un article 1 qui satisfait tout le monde. Sa nouvelle rédaction ouvre à l'ensemble des exploitations, quelle que soit leur forme sociétaire, la possibilité d'acheter les terres qu'elles louent

Lesdites sociétés pourront faire valoir leur droit de préemption, dès lors qu'elles jouissent d'un bail conformément au statut du fermage. Les terres qui n'ont pas été louées avant le 1 janvier 2016 devront, lorsqu'elles seront acquises, être portées par une société distincte. Cela me semble être une bonne solution, qui permettra à ce texte d'être adopté avant la fin de la session parlementaire et donc d'entrer plus rapidement en application. Sur le volet du biocontrôle, l'enjeu principal du combat contre les produits nocifs pour la santé en matière agricole est de trouver

pour garantir une indépendance alimentaire pérenne, ainsi qu'une économie agricole viable. Les solutions réalistes proposées et adoptées par le Sénat ont été conservées. Je m'en félicite. Concernant les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques,

Sur le fond, il était primordial de pouvoir adopter de nouveau les dispositions relatives à l'accaparement des terres agricoles qui avaient été annulées pour des raisons de procédure par le Conseil constitutionnel.

Concernant les produits de biocontrôle et le rétablissement des certificats d'économie de produits phytosanitaires, la

à accélérer la mise en place des nouvelles procédures prévues par la loi d'avenir concernant l'autorisation des produits de biocontrôle et des préparations naturelles peu préoccupantes.

le foncier agricole et le développement de techniques alternatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Je me réjouis, avec les membres du groupe Les Républicains, de l'accord trouvé en commission mixte paritaire la semaine dernière. Je salue le travail et l'implication de notre rapporteur, Daniel Gremillet, qui avait réécrit l'ensemble des dispositions foncières reprises dans cette proposition de loi dès le projet de loi Sapin II.

Ce travail devra être fait dans les prochains mois. En attendant, ce texte complète notre arsenal juridique dans l'objectif de mieux maîtriser le foncier agricole.

à l'acquisition de parts sociales lors des cessions partielles, afin d'éviter, comme ce fut le cas pour l'acquisition des 1 600 hectares de terres dans le Berry par des investisseurs chinois, qu'elles ne puissent pas avoir un droit de regard sur le dossier. part, le texte prévoit l'obligation de passer par une société de portage foncier pour acquérir des terres agricoles. Le Sénat a souhaité exempter de cette obligation l'ensemble des sociétés agricoles, dès lors qu'elles sont locataires des terres qu'elles veulent acquérir et qui sont support de leur activité. Ces sociétés peuvent ainsi faire valoir le droit de préemption du preneur en place. Les députés, quant à eux, craignaient un contournement de la règle avec des baux de complaisance. Un compromis a donc été trouvé, en limitant l'exonération de cette obligation aux baux conclus avant le 1 janvier 2016. Concernant les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, j'avais exprimé quelques doutes et je m'inscrivais dans la logique de notre rapporteur, en faveur d'une écologie positive et incitative. a réintroduit le dispositif de sanction des distributeurs, mais a prévu en contrepartie un bilan à mi-parcours en 2020.

J'en viens aux buis et, plus généralement, aux plantes touchées par des maladies pour lesquelles aucun traitement alternatif aux produits phytosanitaires n'existe. L'accord entre les députés et les sénateurs va dans le bon sens.

Pour autant, il apparaît que le droit actuel permet aux propriétaires privés de parcs et jardins de recourir à des prestataires disposant d'un agrément et du certificat individuel de produits phytopharmaceutiques, même nature. Les mesures sur le biocontrôle posaient question, mais le bilan demandé à mi-parcours sur les CEPP permettra de faire le point et de maintenir le dialogue avec les parties prenantes. Sur le volet foncier, les membres de la majorité sénatoriale ont été à l'oeuvre pour trouver les solutions juridiques à un problème qui est loin d'être anecdotique.

Je reviendrai rapidement sur les dispositifs adoptés, en les replaçant dans le contexte plus large des grandes mutations de nos agricultures. L'accord trouvé sur la mise en oeuvre des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques est à souligner, parce qu'il traduit un progrès, et, plus significativement, une maturité certaine dans l'approche de la question sanitaire en agriculture. La pression sociétale pour une alimentation saine et de qualité justifie pleinement ces dispositions. Je salue le travail du ministre, qui a engagé, avec la loi d'avenir

La dynamique de création de dispositifs alternatifs est bien enclenchée, par les acteurs de terrain eux-mêmes. Il faut s'en réjouir. Je note aussi que, à l'échelon européen, les choses bougent dans le bon sens ; M. le ministre l'a indiqué. Hier, par son vote, le Parlement européen a appelé à un mécanisme simplifié d'autorisation de mise sur marché, plus rapide et plus facile, des pesticides biologiques à faible risque et des produits de biocontrôle. Cette filière doit se développer comme une alternative efficace aux produits phytopharmaceutiques. Compte tenu des enjeux de santé évidents- je pense aux perturbateurs endocriniens -et des risques encourus, y compris pour les agriculteurs eux-mêmes, je souhaite qu'une nouvelle législation voie rapidement le jour, afin d'accélérer les procédures d'évaluation, d'autorisation et d'enregistrement des pesticides à faibles risques. Pour ce qui est de notre texte, et en attendant la généralisation du biocontrôle, je persiste à penser que l'agriculteur ne doit pas supporter seul la responsabilité de l'emploi des produits phytopharmaceutiques. Comme pour la valeur ajoutée agricole ou agroalimentaire, dont on sait qu'elle est trop souvent trop trop faible pour le producteur et qu'elle devrait en conséquence être redistribuée plus équitablement sur toute la chaîne de valeur, la responsabilité de réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques doit être répartie de l'amont à l'aval, des fournisseurs d'intrants aux metteurs en marché. Le texte va dans ce sens. Il faudra veiller à ce que son esprit ne soit pas détourné en pratique au détriment de l'agriculteur. En première lecture, j'avais posé la question de la maîtrise du foncier agricole de notre pays comme un enjeu de souveraineté nationale. Le dispositif que nous avons adopté et que la commission mixte paritaire nous a permis de sécuriser juridiquement aide à faire un grand pas dans ce sens. C'est un point de progrès notable, qui doit nous engager maintenant vers une nouvelle étape, sous la forme d'une loi foncière spécifique qui traiterait du foncier agricole en lien avec l'ensemble du foncier national. Entre autres questions, la capacité financière des SAFER à intervenir efficacement et la rémunération des externalités positives des espaces ruraux et agricoles-

Pour ce qui est du pouvoir d'intervention des SAFER, les moyens nécessaires doivent être disponibles pour que la mission que nous leur confions et que nous avons renforcée avec ce texte puisse être correctement exercée. je propose que le Parlement appréhende la problématique des moyens nécessaires aux SAFER en prenant en compte la réalité des missions, du fonctionnement et des résultats constatés de tous les opérateurs publics du territoire- je pense en particulier aux établissements publics fonciers -qui prélèvent, par la fiscalité directe, des ressources sur les territoires ruraux agricoles qui, en retour, n'en bénéficient pas ou très peu. Au coeur de la loi foncière dont nous pourrions être amenés à débattre prochainement devrait donc figurer l'objectif d'égalité territoriale, de justice territoriale. territoriale, de justice territoriale. Les deux sujets de ce texte nous rappellent que l'agriculture se situe dans un moment de mutation profonde et accélérée. Cela appelle de notre part à tous un bon diagnostic, une problématisation juste et un plan d'action tout aussi pertinent qu'efficient.

À cet égard, l'année 2017 sera essentielle pour l'avenir du modèle de politique agricole commune. Je souhaite que la France fasse valoir l'intérêt de ses paysans et de ses territoires dans le concert agricole européen.

l'un des rapporteurs. Notre agriculture est confrontée, à l'échelon national comme européen, à des défis de sécurité et de qualité alimentaire, des défis économiques, environnementaux, territoriaux et de résilience à l'égard des nombreux aléas dont elle est en permanence l'objet. Pour répondre à ces défis, nous devons faire une analyse juste du fonctionnement de la PAC actuelle et en déduire les objectifs pertinents pour la prochaine, en cours de préparation. La PAC des années 2020 doit être construite sur les objectifs suivants : la garantie de la croissance, de l'emploi et de la compétitivité, la contribution aux enjeux climatiques et environnementaux, le développement de la ruralité, la gestion des risques de toute nature pour une agriculture plus résiliente et plus durable, respect et la prise en compte de la diversité des modèles et l'octroi de soutiens proportionnés. Sans rentrer dans les détails, l'enjeu de gestion et de couverture des risques économiques, la question du niveau et de la garantie du revenu du producteur agricole

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12 du règlement, le Sénat lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte

appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi qu'il nous revient d'adopter définitivement cet après-midi comporte plusieurs dispositions importantes pour le fonctionnement de notre système électrique et gazier. Ses objectifs sont largement partagés, comme en atteste l'accord auquel nous sommes parvenus avec nos collègues députés lors de la commission mixte paritaire du 1 février dernier. En premier lieu, le texte fixe un cadre légal à l'autoconsommation d'électricité. C'était d'autant plus nécessaire que cette pratique est appelée à se développer et qu'elle n'est pas sans conséquence sur les réseaux. Il convenait donc d'en définir précisément les contours. Ainsi, sur l'initiative du Sénat, il a été précisé, d'une part, que l'autoconsommation individuelle devait être limitée à « un même site », afin d'éviter des effets d'aubaine sans bénéfice pour les réseaux, et, d'autre part, que l'autoconsommation collective pouvait s'étendre à tous les à tous les départs basse tension d'un même poste de transformation de moyenne en basse tension. Ce point, qui peut paraître très technique, n'en était pas moins essentiel pour permettre des échanges vertueux d'énergie entre bâtiments résidentiels et tertiaires. De même, le Sénat a clarifié le droit applicable aux petits autoconsommateurs en matière d'exonérations de contribution au service public de l'électricité, ou CSPE, et de taxes locales sur l'électricité. En deuxième lieu, le projet de loi permet d'organiser la traçabilité de l'électricité verte subventionnée par la mise aux enchères, par et au bénéfice de l'État, des garanties d'origines associées à cette production. Un tel mécanisme, introduit à l'Assemblée nationale, empêchera la double rémunération des producteurs et dégagera des recettes qui viendront en déduction des subventions versées aux énergies renouvelables. Pour mieux répondre aux demandes en faveur d'un mix diversifié et d'une énergie produite localement, le Sénat l'a complété de la possibilité de constituer des lots par filière et par zone géographique. Nous avons aussi prévu la faculté pour l'État de n'émettre qu'une partie des garanties, afin d'optimiser les coûts de gestion du système. En troisième lieu, ce texte aborde la question des coûts de raccordement des installations d'énergies renouvelables. Pour faciliter la réalisation des projets les plus éloignés du réseau, le projet de loi rétablit la « réfaction tarifaire » au bénéfice des producteurs, c'est-à-dire la prise en charge par la collectivité d'une partie des coûts de raccordement. Trois précisions importantes ont été apportées au cours de la navette. sur l'initiative de l'Assemblée nationale, la possibilité de moduler le taux de la réfaction selon les filières et la taille des installations a été explicitement prévue. L'aide sera ainsi concentrée sur les plus petits projets, comme l'installation de panneaux solaires sur des bâtiments agricoles. Ensuite, sur la proposition du Sénat, il a été décidé de plafonner le taux maximal de réfaction à 40 % des coûts, ce qui, combiné à la modulation, permettra de réduire la charge de trésorerie pour les entreprises locales de distribution, les ELD ; c'était là un point de vigilance essentiel pour un grand nombre d'entre nous. C'est très clair nous avons réaffirmé le rôle des autorités organisatrices de la distribution d'électricité, aux côtés des gestionnaires de réseaux, dans la maîtrise d'ouvrage des travaux de raccordement. J'ajoute que nos collègues députés ont opportunément élargi le principe de la réfaction aux installations produisant du gaz renouvelable. Cela favorisera l'émergence de cette filière naissante.

le Sénat a enrichi le texte, d'abord en prévoyant la couverture par les tarifs d'utilisation des réseaux des coûts de conversion des sites de stockage, ensuite en actant la nécessité d'un accompagnement des consommateurs aux revenus modestes qui auraient à remplacer un équipement inadaptable, pour lequel le Gouvernement doit maintenant travailler à un dispositif opérationnel, ce à quoi il s'est engagé devant nous. Madame la ministre, vous avez soumis un premier projet au Conseil d'État, qui ne l'a

Pour répondre à cette préoccupation, de nombreuses initiatives ont été prises ces derniers mois dans différents textes, mais une seule a perduré : l'article 86 de la loi de

en réalité que peu ou pas d'effets. C'est la raison pour laquelle le Sénat a proposé d'aller plus loin, en dispensant de règles administratives les anciens moulins équipés pour produire de l'électricité.

car le principe de la dispense des règles applicables aux moulins existants, déjà équipés aujourd'hui ou qui pourraient l'être demain pour produire de l'électricité, a été maintenu.

n'en limite pas la portée pratique, puisque ce sont en réalité les seuls à être concernés par le risque d'« effacement ». Pour éclairer le sujet, je m'appuierai sur quelques données chiffrées. Sur les 19 000 seuils de moulins recensés en France, 15 800 environ sont situés sur des cours d'eau prioritaires, dont 10 000 sur des cours d'eau classés en « liste 1 » et 5 800 en « liste 2 Le classement en liste 1 attestant le très bon état écologique des cours d'eau concernés, il n'a, par définition, pas d'autre impact que celui de préserver leur état pour l'avenir, c'est-à-dire d'interdire toute construction d'un nouvel ouvrage, ou de subordonner le renouvellement de la concession ou de l'autorisation d'un ouvrage existant à des règles permettant de maintenir ce très bon état, ce qui revient donc ce qui revient donc à ne pas modifier les ouvrages existants. Ainsi, outre le fait qu'il est légitime de conserver des règles pour ces cours d'eau « ultra-prioritaires », les 10 000 moulins

La dispense de règles produira en revanche son plein effet pour les 5 800 ouvrages situés en liste 2, qui étaient jusqu'à présent tenus de réduire leur impact sur la continuité écologique dans les cinq les mesures correctrices requises par l'administration pouvant aller jusqu'à l'arasement des seuils. Désormais, ces règles ne s'appliqueront plus pour tous les ouvrages existants qui sont équipés aujourd'hui, ou qui le seraient demain, pour produire de l'électricité

À raison d'une moyenne de 50 kilowatts de production électrique par moulin, et toutes choses égales par ailleurs, c'est donc un potentiel maximal

C'est pourquoi la solution à laquelle nous sommes parvenus me semble résoudre définitivement la question, de manière pragmatique et avec le souci de la conciliation des différents intérêts en présence. Je vous renouvelle mes remerciements sur ce point, madame la ministre.

texte en l'état. Mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer, dans la tribune d'honneur du Sénat, une délégation de cinq députés du groupe d'amitié Turquie-France de la Grande Assemblée nationale turque, conduite par Mme Serap Yaşar, présidente du groupe d'amitié. La délégation est accompagnée par notre collègue Jacques Mézard, président du groupe interparlementaire d'amitié France-Turquie. Arrivée le 13 février, la délégation est à Paris jusqu'au 16 février, pour une visite d'étude principalement centrée sur notre régime institutionnel. Ce thème a été retenu par nos homologues turcs dans le cadre de la réforme constitutionnelle que la Turquie a engagée. La délégation s'est entretenue hier avec des membres de la commission des affaires européennes, présidée par notre collègue Jean Bizet, sur les relations de la Turquie avec l'Union européenne. Elle a rencontré également plusieurs membres de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, présidée par notre collègue Jean-Pierre Raffarin, afin d'évoquer le rôle de la France et de la Turquie face aux grands enjeux géopolitiques actuels, en particulier le conflit syrien et ses conséquences. Le Sénat français entretient des relations de confiance et d'amitié avec la Grande Assemblée nationale turque, nourries d'échanges sur les grandes questions liées à la situation en Syrie qui nous préoccupe tous, mais aussi sur les liens étroits qui unissent la Turquie à l'Union européenne et le développement de nos partenariats économiques, en particulier dans le domaine des transports et de l'énergie. Mes chers collègues, en votre nom à tous, permettez-moi de souhaiter à nos homologues de la Grande Assemblée nationale turque la plus cordiale bienvenue, ainsi qu'un excellent et fructueux séjour. Nous reprenons

Nous avons passé ensemble de longues heures, de longues journées, de longues nuits, il y dix-huit mois, pour cette discussion parlementaire très intéressante et très fructueuse

à la Programmation pluriannuelle de l'énergie, et à l'accord historique sur le climat obtenu à Paris le 12 décembre 2015, et entré en application le 4 novembre 2016.

ce qui explique, à mon sens, le succès mondial de la mise sur le marché par la France de la première obligation verte souveraine, pour 7 milliards d'euros,

les énergies renouvelables électriques produisent désormais, à la pointe de midi, l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires et contribuent donc à la sécurité de l'alimentation ; l'éolien a progressé de 45 % en 2016 les projets de chaleur renouvelable et de récupération aidés par le Fonds chaleur ont augmenté de près de 30 % ; la filière éolienne compte désormais 15 000 emplois sur le territoire français, soit une augmentation de 30 % depuis 2013, ce qui correspond à 4 000 emplois supplémentaires, et sans doute davantage si l'on compte les sous-traitants. Pour prolonger cette dynamique, l'ordonnance relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables que tend à ratifier l'article 1 du projet de loi qui vous est soumis permet une meilleure intégration des énergies renouvelables au marché et au système électrique, et ce pour trois raisons.

Elle permet de doter la France d'un cadre qui facilite le développement de l'autoconsommation. Ce développement est vertueux pour les énergies renouvelables, les réseaux d'électricité et, bien évidemment, les factures énergétiques. J'ai lancé un appel d'offres, l'été dernier, pour le développement de l'autoconsommation dans les secteurs industriels, tertiaires et agricoles. Les 72 premiers lauréats ont été désignés à la suite de cette procédure, qui a rencontré un très grand succès. Peut-être en avez-vous d'ailleurs quelques exemples dans vos territoires,

en particulier, mais pas seulement, sur les territoires à énergie positive. Cette ordonnance prévoit la définition des opérations d'autoconsommation, l'obligation pour les gestionnaires de réseaux de faciliter l'autoconsommation, ce qui représente une grande avancée, et l'établissement par la Commission de régulation de l'énergie d'une tarification d'usage du réseau adaptée aux installations en autoconsommation. autoconsommation. Je suis très attachée à ce que les tarifs d'usage des réseaux intègrent dès à présent ce nouvel usage qu'est l'autoconsommation, pour en favoriser le développement. Elle prévoit enfin l'exonération de taxes sur l'électricité autoconsommée.

Nous avons donc atteint là l'objectif de garantir que l'électricité bénéficiant des dispositifs de soutien nationaux, qui sont financés par tous les consommateurs, profite bien à l'ensemble des consommateurs, sans que les fournisseurs puissent bénéficier d'une double rémunération indue. Maintenir ce principe de non-cumul est également nécessaire pour sécuriser juridiquement les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables, dont j'ai obtenu la-validation par la Commission européenne les 12 décembre et 10 février dernier.

qui ont été encadrés par le décret du 1 avril 2016, le coût du raccordement se révèle parfois un frein pour les projets d'énergies renouvelables, notamment en milieu rural, loin des réseaux. Il s'agit donc d'une mesure d'équité territoriale.

Je vous annonce d'ailleurs que les conventions de concession d'occupation du domaine public maritime pour les parcs éoliens en mer qui sont lauréats du premier appel d'offres pourront être signées dans les prochains jours. C'est donc une étape majeure qui va ainsi être franchie, pour placer la France à l'avant-garde en matière d'énergies marines. l'article 4 clarifie la gestion de la conversion de la nature du gaz acheminé aux consommateurs dans le nord de la France, du fait de la baisse de la production du champ néerlandais.

je vous informe que je proclamerai dans les prochaines semaines les résultats de l'appel d'offres sur la petite hydroélectricité, avec un lot qui sera spécialement réservé aux anciens moulins.

seulement dans le cadre des territoires à énergie positive, qui sont maintenant 500 sur l'ensemble du pays, mais également pour des projets bien identifiés que vous pourriez repérer sur ces sujets d'autoconsommation. Nous serons à vos côtés pour vous permettre de les faire émerger et de créer

et de limiter par exemple l'impact sur le réseau de distribution. Nous pensons au contraire que ces ordonnances brouillent les enjeux en mélangeant délibérément autoconsommation et autoproduction. L'autoconsommation existe dans notre pays, un mouvement commençant à émerger de façon non négligeable en France. Nous ne pouvons nier qu'un encadrement juridique de cette autoconsommation est nécessaire, mais il y a dans le texte un glissement subtil vers l'autoproduction, puisque ledit autoconsommateur pourra aussi injecter et vendre son surplus de production, sans être l'objet de contraintes et de coûts disproportionnés. Cet autoconsommateur conserve le bénéfice des droits des consommateurs et ne doit pas être qualifié de fournisseur d'énergie à l'occasion d'opérations de vente d'électricité. Il peut recevoir une rémunération, étant entendu que cette dernière doit être calculée à partir de la valeur de cette électricité sur le marché, quand bien même il aurait reçu des aides, puisqu'il s'agit d'énergies renouvelables. Sur l'autoconsommation collective, des logements ou des centres commerciaux pourront ainsi produire leur propre électricité et la vendre. Il y a donc bien, pour nous, volonté délibérée de démanteler un modèle centralisé ayant démontré son efficacité dans le passé, une sorte de retour au début du siècle dernier, qui, sous couvert de transition énergétique, va sans nul doute aboutir à la remise en cause de l'égalité d'accès à l'énergie sur l'ensemble de notre territoire, de l'égalité de traitement des usagers, ainsi que des tarifs réglementés, lesquels sont, il faut le rappeler, une forme de contrepartie à l'acceptation par nos concitoyens du choix de la production nucléaire.

avouez-le, d'un modèle familial d'autoconsommation ... Il s'agit ni plus ni moins que de créer un nouveau marché. Manifestement, nous n'avons pas appris des écueils et des abus du développement du solaire ou encore de l'éolien mauvais choix stratégiques, sans véritable pilotage ni planification, qui ne nous ont pas permis de véritablement diversifier notre mix énergétique. Pourtant, comme nous l'avons encore hier, ici même, avec notre question d'actualité au Gouvernement, nous pensons toujours que EDF, RTE et ERDF doivent être les pivots de la transition énergétique et du développement des énergies renouvelables., renouvelables., les mesures de destruction de ce modèle intégré ne sont que la promotion de la création de nouveaux marchés factices et éphémères. À nos yeux, et nous l'avons dit et répété au cours de cette législature, les marchés et le recours exclusif au secteur privé, avec sa logique de profit à court terme, ne peuvent nous permettre de nous hisser à la hauteur des enjeux de la transition énergétique, qui nécessitent des temps longs et d'importants investissements publics, ni d'avoir un véritable service public national de l'énergie. c'est sans doute toute la philosophie de ces ordonnances : casser la notion même de service public national ! L'autoconsommation promue par les différentes ordonnances remet en cause

Nous avions déjà, lors des débats sur le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, souligné la nécessité de faire de la transition énergétique une priorité réelle de la politique économique et budgétaire de la Nation. Plutôt que d'y consacrer les moyens nécessaires, le Gouvernement et sa majorité ont largement misé sur le soutien à l'initiative privée, en s'inscrivant dans une démarche d'ensemble tendant à la privatisation du secteur de l'énergie renforcement du marché de capacité ; renforcement du marché de l'effacement au profit de monopoles privés ; privatisation du secteur historique de l'hydroélectricité ; soutien financier actif aux opérateurs privés du secteur des énergies renouvelables.

sans que cela réponde à un quelconque objectif d'intérêt général. C'est pourquoi, en toute cohérence avec les positions constantes qui sont les nôtres, nous ne voterons pas ce projet de loi. La parole est à M. Jean-Claude Requier. Madame la merci à tous Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la lutte contre le changement climatique rend impérative la diversification de notre mix énergétique. C'est le sens des engagements adoptés par la France ces dernières années avec l'Accord de Paris et la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. En dépit des obstacles normatifs, économiques et financiers, les investissements dans le secteur des énergies renouvelables montent en puissance et les solutions sont incontestablement de plus en plus compétitives pour certaines filières comme l'éolien et le photovoltaïque. Le contexte international est également favorable, puisqu'il existe une véritable dynamique pour parvenir au respect des objectifs ambitieux qui ont été fixés. Toutefois, gardons à l'esprit que la part des énergies fossiles dans la consommation mondiale reste de 87 % depuis quinze ans, d'après le Centre de recherche international la ratification des deux ordonnances prises sur le fondement de la loi relative à la transition énergétique, le présent projet de loi apporte des garanties pour sécuriser le développement de l'autoconsommation et de la production d'énergies renouvelables. outre à inciter les consommateurs et les entreprises du secteur à investir dans la transition énergétique en levant quelques freins qui demeuraient. S'il est naturel de l'électricité à proximité des lieux de production, la décentralisation énergétique doit être préparée, car elle crée un risque certain pour notre système électrique et pour le réseau. Le recours à des moyens de stockage est inévitable, et l'hydrogène devrait avoir, nous l'espérons, un rôle important à jouer. Les membres du RDSE en sont intimement convaincus. Je salue le travail de notre rapporteur, Ladislas Poniatowski, qui a permis de lever les incertitudes qui subsistaient après l'examen du texte par l'Assemblée nationale. Les modifications adoptées par le Sénat ont été retenues par la commission mixte paritaire, ce dont je me réjouis. Une fois de plus, le bicamérisme a fait la démonstration de son utilité. Ainsi, nous ne pouvons que souscrire à la fixation par le présent texte d'un cadre juridique adapté pour l'autoconsommation, qui fait l'objet d'un réel engouement, y compris dans les territoires ruraux. C'est notamment la dérogation à l'obligation de conclure un contrat de vente avec un tiers pour le surplus d'électricité non consommé. Le texte établit, en outre, un cadre fiscal avantageux, avec la tarification spécifique de l'accès au réseau de distribution pour les petites installations, à savoir le « micro-TURPE », et l'exonération de CSPE et des taxes locales pour la production autoconsommée. De même, il facilite et accompagne la production d'électricité renouvelable par l'extension de la priorité d'appel pour les installations dans les zones non interconnectées, le renforcement de la coordination entre les producteurs et les gestionnaires du réseau, régime spécifique d'indemnisation en cas de retard de raccordement pour les installations d'énergies renouvelables en mer. On peut aussi citer la possibilité de recourir à des formes de mise en concurrence, qui repose sur le dialogue entre l'État et les porteurs de projets présélectionnés à partir de leurs capacités techniques et financières. L'article 3,

comme le prouvent notamment les territoires à énergie positive. Cette mesure présente un rapport coût-avantage intéressant, puisqu'elle aura un faible impact sur le TURPE, le taux maximal de réfaction, modulé selon la puissance ou la filière, étant limité à 40 %, alors que les effets seront très bénéfiques pour les petites installations. Par ailleurs, le texte permet d'assurer la traçabilité de l'électricité verte et d'éviter une double rémunération des producteurs en instaurant un système de mise aux enchères des garanties d'origine de la production d'électricité renouvelable subventionnée, organisé par l'État à son bénéfice. Je terminerai mon propos en évoquant l'article 3 , qui porte sur les moulins à eau contribuant à la production d'énergie renouvelable. La loi Montagne, récemment votée, dispose que la gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, ce qui comprend les moulins. Le Sénat a souhaité aller plus loin, en proposant que les anciens moulins ne soient pas soumis à l'autorisation préfectorale et aux contraintes imposées à l'article L. 214-17 du code de l'environnement et destinées à préserver la continuité écologique des cours d'eau. La rédaction de la CMP clarifie le dispositif, en exonérant les moulins régulièrement installés sur les cours d'eau de la « liste 2 des réglementations correspondantes, c'est-à-dire la gestion, l'entretien et l'équipement selon les règles définies par l'autorité administrative, afin d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Nous sommes donc satisfaits de cette avancée.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voilà donc réunis pour nous prononcer de nouveau sur ce projet de loi, qui a fait l'objet d'un vote favorable en CMP. Dans un climat consensuel, les propositions sénatoriales qui avaient été votées avec l'avis favorable du Gouvernement et de la grande majorité des groupes politiques ont ainsi été reprises par nos collègues députés. C'est donc une loi enrichie par le travail du Sénat et l'Assemblée nationale,

accompagner l'essor des énergies renouvelables, organiser une meilleure traçabilité de l'électricité verte, favoriser le raccordement des projets éloignés des réseaux, enfin, pour assurer le changement de la nature du gaz dans le Nord. Pour

L'article 3 issu des travaux de la CMP vise à trouver un équilibre entre le développement de la microélectricité et la préservation de la biodiversité avec la continuité écologique des cours d'eau.,

cette nouvelle version assouplit les règles pour les moulins à eau équipés existant à la date de la promulgation de la loi et installés sur des cours d'eau classés en « liste 2 Désormais, ces derniers ne seront plus soumis aux obligations définies à l'article L. 214-17 du code de l'environnement, aux termes duquel « tout ouvrage [doit être] géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. » Ainsi, plusieurs milliers de petits ouvrages appartenant à notre patrimoine historique sont concernés par cette mesure et seront donc préservés.

En effet, tous les cours d'eau ainsi classés sont loin de présenter les caractéristiques retenues, à savoir une qualité écologique et une richesse biologique particulièrement importantes réclamant une protection administrative renforcée. On peut également s'interroger sur l'intérêt d'intégrer à cette « liste 1 » des cours d'eau considérés comme « réservoirs biologiques », dont la définition est parfois appliquée par l'administration de manière très extensive, sans qu'y soit nécessairement attaché un intérêt environnemental majeur et avéré. Il serait donc opportun, madame la ministre, d'engager à l'avenir une révision-actualisation de cette liste pour l'appliquer aux cours d'eau en très bon état et aux axes migratoires amphihalins durables, qui sont en général des rivières ou tronçons de faible longueur ou situés en tête de bassin.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, comme nous l'avons dit lors de la discussion générale, ce projet de loi est de bonne facture. Sans entrer dans le détail, permettez-moi d'évoquer deux ou trois points forts de ce texte. 1, dont l'objet est de ratifier des ordonnances qui devraient faciliter l'approche des différents maîtres d'ouvrage, sachant que la transition énergétique, c'est aussi une transition intellectuelle et une transition d'usage. Or, les transitions intellectuelles n'étant pas forcément les plus naturelles, autant les inciter, les faciliter et les accompagner. Lors de la discussion générale, à ce sujet, presque tout a été dit,

de la démarche, en revenant sur une notion qui taquine certains d'entre nous et qui provoque, chez le président Lenoir, une très grande méfiance, voire une opposition farouche : je veux parler, bien entendu, de la notion « d'autonomie énergétique pour un territoire. je sais que ce sujet a été évoqué lors de votre entretien avec M. le préfet Carenco, en passe de devenir le « grand chef » de la CRE,

mais je ne pense pas trahir l'esprit de la loi de transition énergétique ni celui de la démarche « Territoires à énergie positive » en réaffirmant que l'autonomie n'est ni la sécession, ni l'indépendance, ni l'isolationnisme, encore moins le divorce ou la séparation. s'agit simplement de souhaiter qu'un territoire, dans une démarche de diversification énergétique, produise plus ou autant que ce qu'il consomme, et ce avec des maîtres d'ouvrage multiples et variés. C'est vrai, il peut travailler en boucle, comme certains l'ont évoqué en commission, mais il reste lié au grand réseau national, dont il a besoin ou qu'il peut alimenter. la véritable transition énergétique, en dehors des pourcentages de nucléaire à telle ou telle date, c'est avant tout une dynamique collective, avec des initiatives citoyennes, industrielles ou militantes. Et l'autoconsommation entre dans une démarche de facilitation de cette dynamique.

en sachant pertinemment que tous les territoires ne seront pas à énergie positive avec un véritable mix énergétique. Vous le savez, faire de l'hydroélectrique dans la plaine des Flandres n'est pas une évidence. Pourtant, de l'eau, d'évoquer la notion de territoire, puisque nous avons voté, à l'unanimité, avant la COP 21, une résolution rappelant qu'il fallait se fonder, pour lutter contre le réchauffement climatique, sur les territoires et les collectivités. La dynamique territoriale est essentielle. Prenez le mot « autonomie » sous la notion de capacité, plutôt que sous celle d'indépendance. J'en arrive enfin à l'article 3 ,

avoir fréquenté pendant une décennie une agence de l'eau, je peux vous le dire, j'en ai vu des gens qui « se battaient contre les moulins », mais j'en ai vu encore plus qui les défendaient au nom du patrimoine et au nom de l'énergie ! Très honnêtement,

Face aux problèmes liés au dérèglement climatique, vous avez voulu, madame la ministre, bâtir un nouveau modèle énergétique, et nous vous avons suivie dans cette voie. Il nous fallait, en effet, agir en responsabilité par rapport au présent et à l'avenir. C'est là un défi gigantesque que nous nous sommes imposé

Concernant l'article 2 et l'interdiction de la valorisation des garanties d'origine de la production d'électricité renouvelable bénéficiant déjà d'un dispositif de soutien public, il n'y a pas de désaccord entre nous. Il s'agit, en effet, d'éviter que le consommateur ne paie deux fois pour la même électricité renouvelable. Il s'agit aussi d'encourager le développement de nouvelles capacités renouvelables directement sur le marché. Concernant le registre des garanties d'origine, j'ai en effet souhaité préciser par voie d'amendement que l'obligation d'inscription sur ce registre ne concernait que les installations produisant de l'électricité à partir d'énergies renouvelables et non pas d'autres installations elles aussi susceptibles de bénéficier d'un bénéfice de soutien. L'article 3, quant à lui, porte sur l'élargissement du bénéfice de réfaction tarifaire pour le raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables. Je le répète volontiers, cette mesure va dans le bon sens, car les coûts de raccordements constituent souvent un obstacle à l'implantation d'installations d'énergies renouvelables. Par ailleurs, et dès lors que l'on considérait que les utilisateurs du réseau devaient bénéficier des mêmes droits, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement, nous avons proposé, un amendement, de donner une base législative

à juste raison, à en soumettre le modèle au comité du système de la distribution publique d'électricité. Je formulerai toutefois une remarque concernant les dispositions relatives à la modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux par les gestionnaires de ces réseaux. Certes, nous saluons l'amendement adopté en séance sur proposition du Gouvernement. à donner la possibilité au gestionnaire de réseau de transport de gaz de conclure, avec des opérateurs de stockage souterrains, des contrats prévoyant la compensation par le gestionnaire du réseau de transport des coûts induits par l'opérateur de stockage par la modification de la nature du gaz. gaz. Nous aurions cependant apprécié qu'une solution soit également proposée par le Gouvernement en faveur des ménages concernés par le changement de gaz.

de crainte de se voir opposer l'irrecevabilité financière. Dès lors, nous nous sommes ralliés, monsieur le rapporteur, à l'amendement par lequel vous proposiez que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur les solutions susceptibles d'être apportées Enfin, nous avons fait adopter un amendement qui vise, en conformité avec le droit européen, à encadrer plus strictement les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut permettre la poursuite d'activité temporaire d'une installation fonctionnant sans autorisation environnementale requise. La poursuite d'activité n'étant possible que le temps de la régularisation de la situation administrative de l'installation, nous avons proposé, et cela fut adopté par le Sénat, que ce délai de régularisation ne puisse dépasser un an. Pour conclure, je dirai que ce texte constitue un pas de plus permettant d'atteindre les objectifs de la loi relative à la transition énergétique. L'ensemble des dispositions législatives de ce texte conforte la volonté politique du Gouvernement de doper le développement des énergies renouvelables en facilitant leur intégration au marché, tout en favorisant cette autoconsommation, qui répond véritablement à une attente sociétale. La prise de conscience écologique renforcera enfin cette dynamique permettant de promouvoir des solutions innovantes. Bien évidemment, madame la ministre, nous voterons ce texte !

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce projet de loi, qui vise à ratifier deux ordonnances relatives à l'autoconsommation d'électricité et à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et qui prévoit des dispositions concernant les réseaux d'électricité et de gaz, s'inscrit bien dans la continuité de la loi relative à la transition énergétique et permet d'en renforcer l'efficacité.

La loi qui abordait la notion d'autoconsommation prévoyait que le Gouvernement prenne une ordonnance pour en définir le cadre juridique.

Ces nouvelles mesures prévoient notamment une définition des opérations d'autoconsommation individuelle et collective, une garantie d'accès des installations aux réseaux publics et contribuent ainsi à son développement et à celui des énergies renouvelables. On peut également se réjouir, M. le rapporteur l'a souligné, d'autres dispositions de ce texte, tel que l'élargissement du bénéfice de la réfaction tarifaire aux producteurs d'électricité renouvelable et de gaz. Celles-ci faciliteront l'implantation d'installations d'énergies renouvelables en milieu rural. D'autres mesures importantes prennent particulièrement en compte la situation d'approvisionnement des consommateurs des consommateurs de gaz dans le Nord- c'est la raison pour laquelle j'y suis sensible. En effet, le gaz distribué dans cette région, en provenance des Pays-Bas, se caractérise par un faible pouvoir calorifique. Cependant, le gouvernement néerlandais a décidé de ralentir l'extraction de gaz naturel du gisement, donc de ne pas renouveler les contrats d'approvisionnement avec la France à compter de 2019.

dans des conditions optimales, la conversion et l'adaptation des installations liées à la modification de la nature du gaz acheminé dans le Nord. Quelque 1,3 million de foyers sont concernés et certains

un rapport indiquant les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour accompagner les personnes aux revenus modestes qui seraient contraintes de remplacer leurs équipements inadaptables au nouveau gaz. Si ces différentes dispositions ont fait l'unanimité dans les deux assemblées, des divergences subsistaient à l'article 3 adopté au Sénat et concernant les

des moulins et les enjeux de la microhydroélectricité, dont on ne peut ignorer l'impact. Enfin, je note que, lundi dernier, la Commission européenne a validé, grâce à votre engagement, madame la ministre, deux régimes d'aides pour le photovoltaïque permettant à la France d'augmenter sa capacité solaire, ainsi qu'un régime de soutien pour l'hydroélectricité. Cette décision contribue à sécuriser le développement des projets d'énergies renouvelables pour la transition énergétique. Pour conclure, nous ne pouvons qu'adhérer aux objectifs de ce texte, qui propose des avancées utiles à chacun et vient appuyer la mise en oeuvre de la loi relative à la transition énergétique et pour la croissance verte. La parole

Qu'il s'agisse de production- tel était l'objet de ce projet de loi -ou d'économies d'énergie, les acteurs locaux et les consommateurs prendront de plus en plus une part active dans la transition énergétique en cours. En donnant à cette transition un cadre légal adapté, celui de la loi de transition énergétique et pour la croissance verte, vous avez, madame la ministre, remarquablement orienté la politique énergétique de notre pays, ce dont je tenais à vous remercier. J'ai pu mesurer aussi sur le terrain votre attachement à donner aux acteurs impliqués les moyens de la réussite. Je me réjouis du succès des territoires à énergie positive et du déploiement des plateformes de rénovation énergétique, autant d'éléments qui profiteront à de nombreux Français. L'atteinte des objectifs fixés pour notre pays passera aussi par la continuité de l'attitude de l'État à leur égard. De très nombreux territoires, leurs maires et les présidents de leurs intercommunalités se sont déjà fortement engagés auprès de leurs populations. Il ne faudra pas les décevoir, et je souhaite vivement que les engagements- financiers, en particulier -pris auprès d'eux soient respectés. Les sujets abordés dans les débats que nous avons eus sur ce texte nous ont permis de nous projeter dans un avenir pas forcément très lointain. Dans cette perspective, la place prise par les productions d'énergies renouvelables et le développement des systèmes locaux de production obligent les législateurs que nous sommes à anticiper le monde énergétique qui vient. France stratégie nous y invite dans une note récente, et la place que devront prendre les collectivités territoriales dans le nouveau contexte doit être repensée. De plus, dans le cadre du marché intérieur de l'électricité, la Commission européenne nous oblige maintenant à traduire dans notre droit national de nombreuses propositions législatives regroupées sous l'appellation de « paquet énergie propre ». À ce stade, deux points de principe retiennent mon attention, la péréquation tarifaire et le devenir des tarifs réglementés. Le développement des énergies renouvelables et des systèmes d'autoconsommation amorce la transition de notre modèle national de gestion de l'énergie électrique. Progressivement, nous allons nous éloigner du modèle centralisé que nous connaissions jusqu'ici pour nous approcher d'un système mixte, décentralisé en partie, voire en totalité, si tel est le souhait. Ce mouvement nous oblige à penser sur des bases nouvelles la question de la péréquation tarifaire, qui est, on le sait, une forme de traduction de l'égalité territoriale à laquelle nous sommes ici tous attachés. Le second point, la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, l'évoque en filigrane dans sa note de problématique relative à la transposition du paquet énergie propre. pose la question importante « de la protection des consommateurs particuliers et résidentiels face à un type d'offre qui pourrait les exposer à des variations considérables à court terme des prix de gros Nous reprendrons ces sujets lors de la discussion des propositions du « paquet énergie propre ». Je souhaite, à titre personnel, qu'il se dégage à la Haute Assemblée un consensus à propos des mécanismes de protection des consommateurs et que les tarifs réglementés soient préservés comme un choix supplémentaire, en application du principe de subsidiarité.

la péréquation tarifaire fait partie de l'héritage de la Résistance et traduit une volonté de solidarité.

je veux redire qu'il est essentiel. M. Poher a apporté des précisions sur la façon dont il voit l'autonomie des territoires. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, sinon que d'autres représentants des territoires clament haut et fort que l'autonomie, c'est tout simplement

par la commission mixte paritaire. Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12 du règlement, le Sénat lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte

bien sûr très largement ce texte, qui concerne la production d'électricité et les énergies renouvelables dans le cadre de la transition énergétique. Ce projet

sur le succès de la COP 21, donc sur l'accord de Paris. Madame la ministre, au nom du groupe socialiste et républicain, nous tenions à vous adresser ici un grand merci ! La parole est

L'ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, visant à préserver l'éthique du sport,

une méthode et une détermination. La méthode a été celle de la concertation. En octobre 2015,

première étape était féconde et réussie. Toutefois, il ne fallait pas pour autant que le riche rapport qui m'avait été remis en avril 2016 reste lettre morte. D'où la seconde étape : la détermination. Il a fallu, dans un délai restreint, élaborer un texte équilibré et porteur de sens, un texte qui offre, aujourd'hui, des avancées considérables au sport français. Bien sûr, rien n'aurait été possible sans la détermination et la ténacité des sénateurs Dominique Bailly et Didier Guillaume, qui ont porté cette proposition de loi dans cet hémicycle,

qui ont su créer les conditions d'un débat constructif au cours de l'examen de ce texte en commission, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. À l'occasion de ce vote, il est important de rappeler que le sport rassemble au-delà des clivages politiques. Vous avez su le montrer une nouvelle fois, et c'est pourquoi je souhaite également saluer le travail collectif mené par l'ensemble des groupes parlementaires, en particulier par Jean-Jacques Lozach, Michel Savin, Mireille Jouve, Claude Kern et Christine Prunaud.

En effet, après la loi du 27 novembre 2015 sur le statut des sportifs, la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, qui a notamment permis la retranscription définitive du troisième code mondial antidopage, la loi du 10 mai 2016 sur les supporters, nous avons l'occasion d'inscrire aujourd'hui une nouvelle ligne, et non des moindres, à notre palmarès. toutefois conscients que notre travail n'est qu'une étape. En effet, demain déjà, il nous faudra trouver de nouvelles solutions pour que le sport que nous souhaitons promouvoir puisse triompher.

de nouveaux instruments pour le contrôle des clubs et un encadrement plus efficace de l'activité des agents sportifs, ainsi que de nouveaux outils en faveur de la transparence, notamment en ce qui concerne les dirigeants des organisations sportives. de nouvelles conditions d'incompatibilité pour exercer dans le monde du sport. Elle permet aussi de nouveaux accords professionnels, afin de lutter contre la diffusion illicite sur internet de contenus sportifs. Une nouvelle instance de réflexion et de conseil permettra de développer le sport féminin et de mieux valoriser celles qui peinent, aujourd'hui, à exercer leur métier de sportives dans de bonnes conditions. De nouveaux dispositifs sont mis en place, à la hauteur des ambitions du sport professionnel français. Ainsi, des garanties d'emprunt pourront désormais être accordées par les collectivités territoriales. On peut également mentionner la sécurisation dans la durée des relations entre les sociétés sportives et leurs associations-supports. Je pense, enfin, aux contrats d'exploitation commerciale de l'image des sportifs professionnels, qui vont permettre aux acteurs de bénéficier d'un dispositif transparent et encadré, tout en donnant un rôle majeur aux partenaires sociaux. Mesdames, messieurs les sénateurs, nous pouvons être fiers d'avoir servi le sport, ses acteurs, ses champions et, à travers cette proposition de loi, tous ses pratiquants. fiers, aussi, d'avoir contribué modestement à nourrir notre rêve olympique commun, celui de « Paris 2024 », qui grandit à mesure qu'approche l'échéance du 13 septembre 2017. l'espère, vous adopterez ce texte dans quelques instants, je m'exprime pour la dernière fois à cette tribune en tant que secrétaire d'État chargé des sports. J'en profite donc pour vous dire, une dernière fois, l'honneur qui a été le mien d'avoir pu penser le sport de demain avec ambition. Je vous remercie très sincèrement d'y avoir contribué.

formulées par le Sénat dans plusieurs rapports publiés ces dernières années et, d'autre part, à servir de support pour mettre en oeuvre certaines préconisations

Cette proposition de loi ne pourra être définitivement adoptée, compte tenu du calendrier parlementaire et de la suspension des travaux en séance publique à compter de la fin de ce mois, que si un consensus se dessine, permettant d'aboutir, aujourd'hui même, à un vote conforme du Sénat. À l'issue de l'examen de la proposition de loi par l'Assemblée nationale, la question qui se pose est donc de savoir si les grands équilibres de cette proposition de loi ont été préservés par nos collègues députés et si le Sénat est en mesure de l'adopter définitivement. L'examen des modifications adoptées par l'Assemblée nationale permet, me semble-t-il, d'apporter toutes les assurances nécessaires. Non seulement les grands équilibres de la proposition de loi

une convention de présentation concernant les agents sportifs qui encadre plus étroitement le dispositif adopté par le Sénat. L'agent sportif ressortissant de l'Union européenne ne pourra, par exemple, recourir à

J'observe, ensuite, que les modifications adoptées à l'article 6, relatif au numéro d'affiliation, qui prévoient que l'association en reste détentrice, constituent un compromis satisfaisant avec la position du Sénat.

que nous ne pouvons que souscrire aux apports de l'Assemblée nationale, qui a prévu que le plafond de la redevance devait être fixé par une convention ou un accord collectif national conclu par discipline, et que le bénéfice de cette redevance serait conditionné

Enfin, l'Assemblée nationale a modifié l'article 12, relatif à un accord professionnel pour lutter contre la diffusion sans droit de contenus sportifs sur internet. Elle a rendu l'accord facultatif, la démarche vertueuse est préservée, ce qui était l'essentiel dans le cadre d'une démarche de droit souple. J'en viens maintenant aux douze articles additionnels adoptés par l'Assemblée nationale. L'ajout de ces nouvelles dispositions illustre l'intérêt que nos collègues députés ont porté à ce texte lors de son examen. Ces articles sont d'importance inégale, même si la plupart constituent des apports importants et judicieux. Mes chers collègues, j'attire plus particulièrement votre attention sur l'article 2 , qui qui encadre le pouvoir réglementaire de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, l'ARJEL, et lui confie un pouvoir de police administrative. À l'article 3 A, ont adopté le principe d'un rapport, à remettre avant le 31 décembre 2017, sur la création d'un délit de fraude mécanique et technologique dans le sport et sur l'élargissement des compétences de l'Agence

L'Assemblée nationale a, par ailleurs, prévu à l'article 6 un rapport sur l'opportunité pour les centres de formation des clubs de bénéficier du régime de financement des centres de formation des apprentis. Cela aussi me semble L'article 13 précise quant à lui le rôle des fédérations concernant les modalités d'accès au sport de haut niveau définies par l'article L. 131-15 du code du sport. Enfin, l'article 15 prévoit prévoit que l'article 3, qui établit une interdiction de parier dans sa propre discipline, entrera en vigueur au 1 janvier 2018. Finalement, les points de désaccord apparaissent donc très limités. Certes, nous regrettons la suppression de

doivent pouvoir financer les infrastructures des clubs en en restant propriétaires, et ceux qui estiment que cette pratique crée un conflit d'intérêts défavorable à l'émancipation du sport professionnel. En proposant de plafonner le montant des subventions dans les stades et les salles de sport utilisés par les clubs professionnels, les signataires de l'amendement déposé au Sénat en première lecture, nos collègues Michel Savin et Claude Kern

Toutefois, pour aboutir, il aurait aussi fallu permettre aux collectivités territoriales d'aider des clubs professionnels à devenir propriétaires de leurs infrastructures, ce qui n'a pas été possible, compte tenu, notamment, de la position du ministère des finances sur ce sujet. La suppression de l'article 7 A ne constitue donc pas, à proprement parler, une surprise. Du moins, notre commission se félicite que la prise de conscience de conscience ait progressé sur la nécessité de faire évoluer le modèle économique du sport professionnel. Hormis cet article 7 aucune disposition essentielle n'a été supprimée par l'Assemblée nationale ; je rappelle en outre qu'aucun des ajouts n'est de nature à nous poser des difficultés C'est donc très naturellement que la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté ce texte

Cet état de fait a conduit à une raréfaction de la diffusion sportive gratuite. Je rappellerai que, voici une quinzaine d'années, certains éditeurs télévisuels avaient tenté le pari de diffuser

fassent l'objet d'initiatives gouvernementales. Cela pourrait se faire, notamment, par le biais d'une modification des décrets liés aux événements d'intérêt majeur ou à l'utilisation de brèves images de sport.

pour exemple la fiscalisation des revenus des transferts de joueurs et des commissions, mais aussi la contractualisation de très jeunes joueurs.

propriétaire de plusieurs clubs de football, qui fait passer les joueurs d'une filiale à l'autre en faussant totalement la donne des transferts.

car le fonctionnement des clubs français s'est toujours fondé sur le principe d'une formation à la pointe, participant à l'éclosion de générations de sélections nationales performantes. De plus, rien n'empêche aujourd'hui un club- ceux-ci sont d'ailleurs nombreux à le faire -d'intégrer des clauses de bonne conduite dans les contrats. Malgré ces réserves, la proposition de loi présente à mes yeux de multiples avancées. de multiples avancées. Je salue notamment le renforcement des missions de la fédération sportive en coordination des ligues professionnelles.

ans après l'arrêt, on avance dans la bonne direction, même si certaines questions restent en suspens.

Au mieux de ses capacités, il a un pouvoir fédérateur, unissant les gens, quels que soient leur origine, leur milieu social, leurs convictions religieuses ou leur situation économique ces mots, prononcés en 2004 par Kofi Annan, alors secrétaire général des Nations unies, à l'occasion de l'année internationale du sport et de l'éducation physique, restent plus que jamais d'actualité. Toutes proportions gardées, bien sûr, c'est ce même état d'esprit collégial qui a animé notre travail sur cette proposition de loi issue de l'initiative de notre rapporteur Dominique Bailly, dont je tiens à saluer ici l'ouverture Associer un membre de chaque groupe politique aux travaux sur ce texte, afin de rechercher, en amont, le consensus le plus large possible, a rendu notre travail non seulement agréable, mais également intéressant et efficace.

Que notre rapporteur se rassure : ces réserves concernent avant tout des modifications adoptées par l'Assemblée nationale ! En effet, si les députés ont amélioré quelques mesures, manière rédactionnelle ou technique, ils ont également introduit des dispositions qui ne m'ont pas toujours paru propices. Vouloir durcir l'accès au métier d'agent sportif, en excluant les personnes condamnées pour fraude fiscale, paraît salutaire eu égard à l'exemplarité et au civisme que l'on peut attendre des agents dans le conseil qu'ils doivent prodiguer aux joueurs. En revanche, s'il était bien nécessaire d'étendre la liste des infractions pour lesquelles une condamnation rend impossible l'accès à la profession d'éducateur sportif, notamment pour tout ce qui concerne les délits de prostitution de mineurs ou de harcèlement sexuel,

que comporte le métier d'éducateur sportif, en particulier dans les quartiers en difficulté, où une expérience de repenti n'est jamais sans effet sur les jeunes.

Notre assemblée gagnerait à se pencher sur le rééquilibrage qu'il faudrait mettre en place entre le sport professionnel et le sport amateur. bien ! Enfin, et c'est là une préoccupation chère à notre groupe, je regrette la suppression de l'article 7 A. Nos collègues députés ont considéré que celui-ci contrevenait à la libre administration des collectivités territoriales et faisait obstacle à de nombreux projets en cours. Je pense, au contraire, que le temps était venu d'adresser un signal concernant la régulation du financement par les collectivités territoriales de nouveaux équipements sportifs. Ces équipements, qui nécessitent de gros investissements, ne donnent lieu qu'à une redevance précaire par nature, puisqu'elle dépend des résultats sportifs du club qui l'occupe. Certes, avec la garantie d'emprunt, il sera possible pour les collectivités locales de soutenir l'investissement sans avoir à sortir de l'argent frais ; il faudra néanmoins, pour que ce soit tenable, que les clubs ne fassent pas défection ensuite. Pour autant, ce texte contient des avancées essentielles et attendues par le monde sportif, avancées qui doivent être validées avant la suspension de nos travaux. La pratique sportive professionnelle est aussi un spectacle sportif qui, ce faisant, met en jeu son image auprès du grand public. Aussi les chartes éthiques et déontologiques dont doivent se doter les fédérations viendront-elles préserver et protéger les valeurs du sport médiatisées lors de ces représentations. De la même manière, les déclarations de situations patrimoniales et d'intérêts des présidents de fédérations sportives délégataires- ne l'oublions pas -renforceront la nécessaire transparence et l'exemplarité dont doivent faire preuve ces fédérations.

Enfin, je me réjouis, en tant que membre de la délégation aux droits des femmes, de la promotion accordée au sport féminin par le biais de la Conférence permanente du sport féminin, qui doit accompagner son développement et sa médiatisation réelle- j'appuie délibérément sur ce dernier mot. Les arguments sont naturellement identiques en ce qui concerne le handisport. Mes chers collègues, dans la continuité de l'esprit collectif qui a animé ce travail, le groupe du RDSE votera à l'unanimité en

Loin des clivages politiques et au service de l'intérêt général, les échanges entre vous, monsieur le secrétaire d'État, et les différents groupes du Sénat ont permis de déboucher en première lecture sur un texte d'équilibre. Quelques semaines plus tard, nous sommes en mesure d'adopter définitivement un texte, qui certes ne constitue pas le « grand soir » de la législation sur le sport, mais qui consacre des avancées attendues par les fédérations et les clubs de sport professionnels. Ces avancées répondent à deux urgences largement reconnues. D'une part, il s'agit de faire évoluer la législation, afin de protéger le sport et les compétitions sportives des risques auxquels ils sont exposés. Violences dans les stades, versements frauduleux, conflits d'intérêts, matchs truqués, dopage sont autant de fléaux qui ruinent l'image du sport professionnel, dont l'esprit est pourtant à mille lieues de ces pratiques.

L'initiative de notre collègue Dominique Bailly était donc nécessaire. Sous son impulsion, en commission- je le remercie de m'avoir étroitement associé aux travaux -, puis en séance, nous avons parfait le dispositif de la proposition de loi, qui nous revient de l'Assemblée nationale pour partie améliorée, pour partie réécrite, voire amputée de certains articles. Parmi les améliorations apportées par l'Assemblée nationale, je tiens à souligner les dispositions en matière de contrôle financier des agents sportifs, notamment l'introduction d'une incompatibilité en cas de condamnation pour fraude fiscale. Mes chers collègues, vous l'avez compris, je regrette que certaines des dispositions que nous avions adoptées aient été modifiées par les députés. J'en prendrai deux exemples, de nature différente.

Le désengagement des collectivités territoriales du financement des installations sportives utilisées par les clubs professionnels est difficilement envisageable tant que ces clubs n'ont pas la capacité de devenir propriétaires de leurs installations, je le reconnais. Néanmoins, cette disposition aurait constitué un signal à l'endroit des clubs. Nous devrons donc travailler dans les prochains moins sur les conditions dans lesquelles ce plafonnement pourrait être envisagé.

pour trouver des solutions concrètes au développement du piratage des programmes audiovisuels sportifs. Je redoute néanmoins l'échec des discussions, qui nous amènerait à légiférer dans plusieurs années, alors que l'urgence est constatée aujourd'hui. Beaucoup reste encore à faire. Si elle n'est pas parfaite, cette proposition de loi constitue toutefois une étape importante pour les ligues et les clubs. C'est la raison pour laquelle le groupe de l'UDI-UC s'engage en faveur d'un vote conforme : il faut que ces dispositions entrent en vigueur au plus tôt. chers collègues, nous nous retrouverons dans les prochains mois pour discuter de mesures tout aussi urgentes, mais sans doute moins consensuelles : à bon entendeur

Si elle ne répond pas à tous les besoins actuels du monde sportif, elle constitue cependant une étape importante en matière de transparence et d'éthique. Le travail des deux assemblées pour permettre l'amélioration d'un texte issu lui-même d'une large concertation- la Grande Conférence sur le sport professionnel

Au chapitre des belles avancées issues de l'Assemblée nationale, notons l'interdiction pour toute personne ayant été condamnée pour fraude fiscale de détenir une licence d'agent sportif. Cette disposition nous semble trouver toute sa légitimité dans un texte ayant notamment pour objectif la transparence des flux financiers dans l'économie du sport.

L'article 3 A ouvre le débat sur la création d'un délit de fraude mécanique et technologique. À l'image des dernières inventions en la matière il nous semble important de réfléchir à la création d'un délit nouveau, mais aussi de définir dans quelles mesures l'AFLD peut être compétente sur cette question. Comme pour les questions relatives au dopage, les différentes formes de tricherie évoluent. Nous devons faire en sorte que notre arsenal législatif évolue également.

Diffusion télévisuelle de programmes nouveaux, événements et tables rondes ont été particulièrement remarqués. La marraine de cette initiative est Gwladys Épangue, double championne du monde et médaillée de bronze olympique de taekwondo, le parrain est Souleymane Cissokho, médaillé de bronze de boxe. le thème choisi est « La médiatisation et la mise en valeur du sport féminin dans les régions »- il n'y a pas que Paris ! Rappelons que ce type de manifestation est essentiel, non seulement pour faire connaître le sport féminin, mais aussi pour inciter les femmes à la pratique du sport et pour permettre au public de suivre des compétitions sportives

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, madame la présidente de la commission de la culture, monsieur le rapporteur, mes chers collègues,

Nos échanges se sont déroulés dans un état d'esprit de qualité et dans une volonté de consensus : nous avons toujours eu le souci de privilégier l'intérêt général. Monsieur le secrétaire d'État, en marge de votre dernière cérémonie de voeux, vous avez insisté sur le fait qu'« une révolution culturelle devait avoir lieu dans le sport professionnel », soulignant cependant que vous n'étiez « ni Nostradamus ni David Copperfield

Nous pouvons cependant la considérer comme la première étape d'un processus qui doit nous amener à réfléchir, en étroite collaboration avec le mouvement sportif, à son avenir, afin de donner à la France les moyens de ses ambitions. texte en première lecture, nous avons adopté des amendements, dont certains ont été supprimés au cours de la navette parlementaire. Nous voulions aller plus loin en matière de financement, avec l'élargissement de la taxe Buffet aux compétitions étrangères diffusées en France dans lesquelles la France est représentée. Cela aurait contribué à rééquilibrer la solidarité entre sport professionnel et sport amateur. En effet, les écarts de financements sont aujourd'hui gigantesques entre les sports très médiatisés et les sports plus « intimistes », qui participent pourtant grandement au rayonnement de la France. Et encore, nous ne parlerons pas ici des différences de financements entre les compétitions masculines et les compétitions féminines. Le modèle de la taxe Buffet est intéressant, mais doit être modernisé ; c'est que nous proposions.

nous avons soumis à votre vote un amendement visant à limiter le financement des dépenses de construction d'une nouvelle enceinte sportive pour les collectivités territoriales, si cette structure est destinée à être utilisée majoritairement par une société sportive. L'établissement d'une réglementation dans ce domaine nous semble nécessaire pour éviter les dérives. Les clubs doivent être encouragés à devenir propriétaires de leurs infrastructures. Supprimée, cette mesure devra être remise sur la table dans un avenir proche. Il nous faudra adapter ses conditions d'application et imaginer une contribution nécessaire du secteur privé dans une proportion minimale, dans le cadre des investissements dans les infrastructures sportives. Nombreux sont les acteurs qui, lors de la première lecture, étaient très sceptiques face à cette disposition. Ils font aujourd'hui le constat qu'elle devra un jour être sérieusement envisagée, afin de protéger nos collectivités, mais aussi nos clubs. L'ouverture des débats à laquelle nous avons contribué est donc une bonne chose pour l'avenir. Cette décision permettra de couper peu à peu le lien, aujourd'hui très fort, mais totalement dépassé, entre collectivités et clubs de sport professionnels. Aujourd'hui, de nombreux points décisifs, défendus par l'ensemble des groupes politiques, sont présents dans ce texte : l'éthique sportive, l'amélioration de la compétitivité des clubs, avec le contrat commercial, la reconnaissance du droit d'usage du numéro d'affiliation, la lutte contre le illégal et la garantie d'emprunt par les collectivités locales, très attendue par certains clubs professionnels, et bien d'autres.

Aujourd'hui, celle-ci est interdite, afin de protéger les collectivités territoriales, mais, nous le voyons bien, la protection de ces dernières passe par l'adoption d'une telle mesure : elle permettra en effet aux clubs d'investir directement et relâchera donc la pression financière sur les collectivités, qui sont aujourd'hui étranglées. Ces dernières n'ont plus les moyens d'investir seules dans des stades ou infrastructures sportives utilisés majoritairement par des clubs professionnels. La modernisation du statut des agents sportifs ressortissants d'un État membre de l'Union européenne est aussi un point essentiel. Bien que cela ne réponde certainement pas à l'ensemble des questions concernant cette profession, il est aujourd'hui plus que nécessaire de le réguler et d'assurer sa transparence, et ce dans l'intérêt premier des sportifs et du sport. Je tiens aussi à mettre en valeur la mesure concernant le numéro d'affiliation. Les investisseurs ont besoin d'une telle garantie, qui doit leur permettre d'assurer à leur investissement, tout en protégeant les associations sportives qui restent les propriétaires de ces numéros d'affiliation. La question tant attendue de la rémunération des sportifs est aussi traitée, avec une distinction désormais possible entre salaire et redevance. Cela doit remettre le sport français dans une dynamique compétitive et renforcer l'attrait du sport professionnel français. L'article 12, que nous avions introduit en première lecture, est lui aussi très important. Il permet d'assurer aux diffuseurs des compétitions sportives une protection contre le piratage illégal de ces contenus, au travers d'un accord professionnel entre les acteurs du milieu. Nous pouvons regretter que l'article ait été modifié par l'Assemblée nationale, ce qui limite sa portée normative, mais l'inscription dans la loi d'une telle mesure est extrêmement importante et pleine de sens elle a vocation à sécuriser les investissements dans le monde du sport, qui contribuent à son développement. La disposition prévue à l'article 12 est fondamentale tant pour les acteurs du monde du sport que pour les diffuseurs TV. Le Sénat aura à coeur de veiller à la mise en oeuvre effective de cette disposition, la lutte contre le fléau du piratage nécessitant la mobilisation de tous les acteurs. Bien d'autres dimensions toutes aussi importantes ont été intégrées au texte : encouragement au développement du sport féminin, en lui assurant une plus grande visibilité, gouvernance, lutte contre le dopage et le trucage des compétitions grâce à la création d'un délit de fraude mécanique, introduction du concept de corruption dans le sport, extension des pouvoirs des DNCG, soutien plus poussé en faveur du handisport, rédaction d'une charte éthique sportive, plus grande régulation plus grande régulation des jeux d'argents liés au sport ou encore promotion du français à travers le monde. Tous ces sujets montrent l'ampleur de la tâche qui nous incombe,

une réflexion plus large sur ces sujets aujourd'hui si importants, car le milieu sportif est en pleine mutation. Alors que Paris et la France connaîtront dans moins de sept mois leur avenir olympique,

Conscients de l'importance de la transparence dans la vie publique, nous avions souhaité élargir aux présidents de fédérations, de ligues, du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français, les obligations de déclaration de situation patrimoniale et de déclaration d'intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Au regard de la mission de service public qui incombe à ces personnalités, il ne me semblait pas excessif d'aligner les obligations déclaratives de ces responsables sur celles des parlementaires et des membres du Gouvernement. La prévention des conflits d'intérêts est un élément crucial et notre initiative place la France parmi les pays disposant des standards les plus exigeants pour atteindre ce but.

L'autorisation faite aux ligues professionnelles de se porter partie civile pour les infractions concernant l'intérêt collectif des clubs ou l'intégrité des compétitions est bienvenue. Il semble en effet logique de considérer que ces structures sont légitimes à bénéficier d'éventuelles réparations, mesure où elles sont directement concernées, l'image de compétiteurs loyaux étant cruciale pour la réputation de ces ligues. Nous en connaissons une éclatante illustration avec le cas du club de handball de Montpellier, qui a été déclaré irrecevable en tant que partie civile dans l'affaire des paris présumés suspects, qui dure depuis maintenant cinq ans. ans. Rappelons que cette affaire, toujours en cours, a provoqué la fuite d'une partie de l'équipe, ainsi que de plusieurs sponsors, affaiblissant considérablement le club. De même, l'extension du droit à la partie civile des ligues pour les violences commises durant des compétitions sportives me semble un progrès certain. Face à des comportements inadmissibles et révoltants, qui présentent une image dégradée et à l'opposé des valeurs que véhicule l'esprit de compétition sport, il semble normal que les ligues, qui cherchent à faire vivre dans les championnats l'éthique du sport, puissent demander réparation. Il s'agit de reconnaître la place naturelle des ligues professionnelles aux côtés des victimes de la violence d'une petite minorité de supporters. Concernant l'article 1 , nous ne pouvons que saluer l'initiative de nos collègues de l'Assemblée nationale d'avoir comblé un vide juridique préoccupant, où plusieurs infractions majeures entraient manifestement en conflit ouvert avec les qualités requises à l'exercice du métier d'éducateur sportif. Dans le cadre du volet visant à renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives, des avancées significatives ont été actées, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Bien qu'il n'y ait pas, à ma connaissance, de cas de fraude technologique répertorié en France en compétition, il n'est pas inutile, me semble-t-il, d'engager la réflexion sur cette question. Comme le disait Mme la rapporteur à l'Assemblée nationale, le sujet n'est certainement « pas assez mûr Toutefois, il est important que nous puissions disposer du rapport qui devra être rendu d'ici à la fin de l'année. Nous devrons être vigilants, afin que ce type de pratique ne sorte pas du domaine de l'anecdotique. Dans le cas contraire, il nous faudra certainement créer de nouveaux délits et peines et confier à l'Agence française de lutte contre le dopage une nouvelle compétence, qui ne manquera pas de soulever de nouvelles exigences concernant la dynamique de son financement.

pour la bonne exécution de ses missions, un pouvoir de police administrative, est atteint. Je rappelle que la Cour des comptes préconisait en 2016 une remise à plat de la régulation des jeux d'argent. De même, afin de lutter contre certaines dérives en matière de manipulation sportive, le rôle des ligues professionnelles concernant l'interdiction de paris sportifs, ainsi que l'étendue de ces interdictions, est particulièrement renforcé. Face à ces difficultés nouvelles, qu'illustre le procès des paris présumés suspects touchant le club de handball de Montpellier et face à la difficulté de détecter de tels comportements, un principe d'interdiction plus général semble une avancée utile pour éloigner le risque de ce type d'infraction. À l'image du dopage, le soupçon même, sans démonstration ou preuve, fait des dégâts considérables sur la réputation de certaines compétitions et érode violemment les valeurs que celles-ci sont censées véhiculer et illustrer.

l'exigence de qualification ou d'expérience professionnelle minimale n'est plus de mise pour le conventionnement, mais le droit européen lui-même va faire passer de deux ans à un an l'expérience des agents sportifs communautaires souhaitant exercer de manière occasionnelle en France. La limitation à une convention sportive par saison est essentielle, pour bien entériner le fait qu'il s'agit d'une dérogation pratique, qui, concrètement, ne touchera que quelques joueurs par an. Les craintes que nous pouvions avoir au regard de la première version du dispositif ne sont plus justifiées grâce à la mise en place de plusieurs garde-fous : la transmission des conventions aux fédérations délégataires, assortie de sanctions en cas de non-respect de cette obligation, ainsi que la nécessité pour l'agent sportif communautaire cocontractant de disposer de l'autorisation d'exercice dans un pays européen. De même, nous pouvons être particulièrement satisfaits de l'introduction d'une disposition excluant de la fonction d'agent sportif les personnes ou structures condamnées pour des faits de fraude fiscale. Ce nouvel article illustre l'équilibre que nous devons définir, entre la souplesse offerte aux clubs pour assurer leur compétitivité et la prise en compte, sans naïveté ou exagération, de certaines pratiques douteuses, bien que très minoritaires. La pose d'une nouvelle pierre dans l'infrastructure du contrôle financier de l'activité des agents sportifs doit également être saluée. Le rôle et les pouvoirs accrus des DNCG, y compris en matière de supervision des achats et cessions de clubs, font avancer la sécurité économique des clubs et des joueurs on s'achemine vers une des solutions les moins contraignantes, tout en étant efficace pour tenter de mettre de la lumière dans les divers flux financiers qui touchent au sport professionnel. Il nous faudra veiller particulièrement au fait que les DNCG puissent remplir parfaitement ces missions nouvelles, qui sont cruciales pour la viabilité économique et financière de certains écosystèmes sportifs brassant beaucoup d'argent. Sur ce point également, nous devrons dresser un bilan dans quelque temps, pour nous assurer de la réussite de ce dispositif de contrôle et, le cas échéant, proposer de nouvelles solutions. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place de contrats commerciaux permettant de rémunérer l'image d'un sportif professionnel, les DNCG seront également destinataires de ces documents pour en favoriser le contrôle. Sur cette initiative, il faut d'ailleurs saluer le travail de réécriture de nos collègues députés. Les risques, soulevés à plusieurs occasions, d'un usage détourné de ces droits à redevance en vue d'une forme d'optimisation sociale sont également contingentés. La définition d'un seuil de rémunération minimale au titre du contrat de travail, ainsi que d'un plafond pour le montant des redevances, est une bonne solution, de même que le renvoi à un accord collectif national ou à une convention collective par discipline. Il me semble effectivement que les écarts importants de rémunération entre les différents sports professionnels rendaient inappropriée une définition monolithique du plafond. Enfin, l'inclusion des URSSAF pour le recouvrement et le contrôle de la contribution sur ces redevances sécurise le dispositif. le plafonnement des subventions des collectivités locales pour les dépenses de construction de nouvelles enceintes sportives, nous avions exprimé notre désaccord. Je suis donc tout à fait rassuré de voir l'Assemblée nationale remettre à plus tard l'introduction d'une telle contrainte. Cela ne signifie pas pour autant que les inquiétudes de fond sur les subventions des collectivités territoriales pour de tels projets ne sont pas justifiées. Toutefois, il nous semble nécessaire de ne pas précipiter l'action avant le temps de la réflexion et d'introduire hâtivement une disposition aux conséquences floues, d'autant plus que celle-ci mettait en péril le principe constitutionnel de libre administration des collectivités. À l'inverse, la garantie d'emprunt des clubs sportifs pour l'acquisition, la réalisation ou la rénovation de leurs équipements sportifs lèvera l'hypothèque qui pesait sur certains projets de premier ordre à travers le pays, comme le projet d'Arena porté par le club de basket de Strasbourg. Il s'agit d'une véritable avancée, qui permettra d'accompagner la transformation progressive du modèle économique des plus grands clubs sportifs de notre pays. Face à la montée en puissance de la diffusion en sur internet des compétitions sportives et à la difficulté de combattre le piratage des contenus sportifs, la possibilité de négocier un accord entre les acteurs du sport professionnel et les diffuseurs permettra une amorce de solution à cette situation.

pouvez-vous nous en dire plus sur le groupe de travail qui doit s'atteler à ce chantier et sur l'éventuel calendrier proposé ?

Par ailleurs, nous nous inscrivons ici dans la continuité de la loi du 1 février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs. Il faudra aller plus loin dans les années qui viennent sur plusieurs sujets importants. Il s'agit notamment des liens entre sport professionnel et sport amateur, une problématique qui transcende la seule répartition des droits télévisuels, la reconnaissance des centres de formation des clubs professionnels, sujet évoqué à l'article 6 ,et de l'amélioration du dialogue social entre les différents acteurs de la filière. Je pense notamment aux observations de la Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs, plus loin sur la transparence des flux financiers générés par les transferts de joueurs et sur la gouvernance du sport professionnel. À cet égard, une mission d'information sénatoriale présentera prochainement ses conclusions dans un secteur circonscrit, celui du football professionnel.

approfondir la question du sport à la télévision et de son accès gratuit, voire réfléchir à l'assouplissement de certains aspects de la loi Évin, afin d'améliorer la compétitivité des clubs.

aux compétitions sportives étrangères ou encore la mise en forme d'un type de contractualisation entre l'État et les fédérations pour favoriser le développement du sport professionnel féminin, n'ont pas été intégrées dans la proposition de loi.

mais également pour le sport en général. En effet, le sport professionnel se doit d'être irréprochable s'il veut être le moteur du développement des pratiques sportives dans notre pays et un facteur de cohésion sociale. La

des recettes fiscales de l'État. En 2009, le dispositif fiscal, qui avait concerné 1 581 sportifs, avait grevé les recettes fiscales de plusieurs dizaines de millions d'euros.

Par ailleurs, les éléments avancés jusqu'à présent, notamment en ce qui concerne l'image des joueurs, ne nous convainquent pas. En effet, les clubs ont depuis longtemps intégré dans les contrats des joueurs un certain nombre de clauses et de dispositions disciplinaires permettant de préserver l'image de l'institution. Je vous remercie,

Le droit à l'image collective voté en 2009 et abandonné en 2010 était une niche fiscale, qui bénéficiait à l'ensemble des joueurs. C'est la raison pour laquelle

explication de vote. On peut être effectivement choqué par le niveau de rémunération de certains sportifs professionnels, en particulier de certains footballeurs,

juste titre, le texte prévoit que les contrats d'image individuelle qui seront signés devront être transmis à la Direction nationale de contrôle de gestion.

une dette annuelle pour la mairie du Mans d'environ 450 000 euros auprès du concessionnaire Le Mans Stadium- si ce chiffre est exact, c'est énorme ! Ce système repose sur le principe de collectivisation des risques et de privatisation des profits.

le rapporteur.

à des élus locaux ou à des dirigeants de club. C'est à travers ce type d'articles que l'on incite les collectivités

travers des articles 13 et 14 adoptés à l'Assemblée nationale sur l'initiative de mon collègue Christophe Premat. L'article 14 indique que les établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger favorisent la pratique sportive de haut niveau. Comme vous le savez, monsieur le secrétaire d'État, l'article L. 331-6 du code de l'éducation dispose que les établissements scolaires du second degré permettent la préparation des élèves en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau, et la pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention. Comme vous le savez également, ces articles du code de l'éducation sont censés s'appliquer aux établissements scolaires français à l'étranger. Malheureusement, dans les faits, des élèves membres du réseau d'enseignement français à l'étranger qui, au vu de leur talent et de leur situation- ils sont membres d'un club sportif de haut niveau pourraient bénéficier du statut du sportif de haut niveau éprouvent des difficultés à s'inscrire à l'option sport de haut niveau au baccalauréat, car leur club ne figure évidemment pas sur les listes ministérielles. Récemment, le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Thierry Mandon, indiquait en réponse à ma question orale sur ce sujet : « Quant Quant à ceux qui pratiqueraient leur discipline dans un club étranger qui ne figure pas sur les listes ministérielles, seule une convention entre la fédération française du sport considéré et le club local pourrait être une solution alternative à la situation actuelle. Aussi, monsieur le secrétaire d'État, je vous serais très reconnaissante de bien vouloir m'indiquer si la signature d'une telle convention est concrètement envisageable et si elle permettra réellement aux élèves du réseau d'enseignement français à l'étranger de s'inscrire à l'option sport de haut niveau au baccalauréat.

voix, dans le texte de la commission, l'ensemble de la proposition de loi visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs. Mes chers

M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d'un sénateur appelé à siéger au sein du conseil de surveillance et de deux sénateurs appelés à siéger au sein du comité stratégique de la Société du canal Seine-Nord Europe. Conformément à l'article 9 du règlement, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a été invitée à présenter des candidatures. Les nominations au sein de ces organismes extraparlementaires auront lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement.

L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant réforme de la prescription en matière pénale

à l'Assemblée nationale par les députés Alain Tourret et Georges Fenech. Tous avaient raison de rappeler que, fondé sur des principes simples fixés pour l'essentiel à l'époque de la codification napoléonienne, le droit de la prescription était entré dans une ère d'instabilité marquée par la multiplication chaotique des dispositions particulières et dérogatoires aux règles classiques du droit. De surcroît, cette évolution, décidée notamment par la chambre criminelle de la Cour de cassation, s'inscrivait dans des perspectives contradictoires selon que l'on envisage le domaine pénal ou civil. En effet, dans le premier cas, les délais tendaient à s'allonger tandis qu'en matière civile, et en dépit de nombreuses nuances, la prescription trentenaire cédait de plus en plus le pas à des délais plus courts. Il fallait donc rétablir une sécurité juridique et la qualité des propositions émises a eu raison de toutes les fatalités. le Parlement a réussi à traiter une question complexe et difficile là où bien des gouvernements avaient échoué. J'ai notamment retrouvé, parmi les multiples projets, le dernier qu'avait conduit la Chancellerie et qui constituait un avant-projet de réforme du code de procédure pénale, soumis à concertation par

Il tend à répondre à l'inadaptation du cadre juridique actuel afin de mieux protéger les intérêts de la société tout entière. Évidemment, l'allongement des délais de prescription de l'action publique de droit commun constitue l'apport le plus important de ce texte

les modalités de computation des délais, toujours source de nombreuses difficultés. Le texte harmonise également les délais de prescription de l'action publique et des peines, ce qui est une disposition importante. Il est sain que le législateur intervienne, car le justiciable, qu'il soit victime ou prévenu, a le droit de savoir selon quelles règles l'action publique sera engagée, et, s'il est condamné, pendant combien de temps la peine pourra être exécutée. Tous les justiciables

En l'adoptant, nous allons nous rapprocher des règles en vigueur dans les pays qui ont maintenu la prescription, puisque certains, notamment les pays anglo-saxons, ont choisi de renoncer à ce principe. Cette évolution intègre aussi le fait que le rapport au temps a changé en France. Il est difficile d'évoquer aujourd'hui le droit à l'oubli, car cette notion n'est plus acceptée : les victimes ne la comprennent pas. Le rapport au temps a aussi changé pour les auteurs présumés de délits et de crimes, qui pensent pouvoir s'abriter derrière des délais courts de prescription. Le rapport au temps a enfin changé avec les progrès de la science, notamment grâce aux recherches de l'ADN et à toutes celles qui sont susceptibles aujourd'hui d'aider au dévoilement de la vérité judiciaire. Il fallait donc en finir avec les acrobaties juridiques auxquelles les magistrats du parquet étaient contraints d'avoir recours pour pouvoir engager des poursuites dans certaines affaires criminelles, dans lesquelles il aurait été incompréhensible que les auteurs des faits ne puissent être poursuivis. Voilà pourquoi le Gouvernement considère que ce texte, dont il n'était pas à l'origine, est utile et précieux. Seule une disposition relative à la loi de 1881 a interdit son adoption par un vote conforme. Il a donc fallu une commission mixte paritaire, qui n'a pu aboutir, ce qui nous vaut le plaisir de nous retrouver aujourd'hui. Le Gouvernement souhaite maintenant que ce texte termine son cheminement. La parole est à M.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme de la discussion de cette proposition de loi, qui est importante. effet, elle modifie le régime de la prescription, qui est l'un des fondements de notre législation pénale, et ce depuis longtemps. La prescription se justifie, traditionnellement, par la difficulté d'administrer la preuve d'un crime ou d'un délit quand un long délai s'est écoulé.

parce qu'elle met en avant la protection des victimes. De ce fait, nous n'avons, hélas ! pas pu obtenir d'accord au sein de la commission mixte paritaire.

passé le délai de trois mois. Voilà où nous en sommes ; voilà la raison pour laquelle notre rapporteur, François-Noël Buffet, qui ne pouvait présenter lui-même les positions de la commission ce soir

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la commission mixte paritaire n'est pas parvenue à élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion

relatives à la prescription de l'action publique, en particulier les articles 7 à 9 du code de procédure pénale, en doublant les délais applicables en matière criminelle et délictuelle. Cette proposition de loi est conforme à la logique dominante de ces derniers temps, durcir toujours davantage la justice pénale. Cette logique est pourtant désapprouvée par de nombreux professionnels du droit. L'article 1 de cette proposition de loi modifie les dispositions relatives à la prescription de l'action publique en doublant les délais applicables en matière criminelle et délictuelle. La commission des lois du Sénat a défendu cette solution en arguant que certaines contraventions sont d'anciens délits requalifiés. Nous l'avons déjà dit lors de la première lecture : il nous paraîtrait plus efficace de revoir l'échelle des peines plutôt que de prolonger les délais de prescription de toutes les contraventions.

Les cas les plus graves, comme les faits délictuels ou criminels que la victime tarde à dénoncer, relèvent dans la majorité des cas de règles de prescription spécifiques et dérogatoires.

respecter la victime sans la faire passer pour responsable de ce qu'elle a subi ; lutter contre la banalisation ; faciliter le recueil du témoignage,

yeux, cette réforme met en péril le droit au procès équitable. Au-delà d'un certain laps de temps, la prescription se veut garante du procès, car le dépérissement des preuves et de la capacité à s'y opposer demeure une réalité.

n'en est qu'une partie mineure -, d'autres moyens que l'allongement de la prescription existent pour améliorer l'aide aux victimes. Je les ai déjà évoqués. Cette proposition de loi aurait dû s'y intéresser plutôt que de s'engouffrer dans une politique pénale toujours plus répressive. C'est la raison principale qui nous conduit

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, au-delà du désaccord spécifique qui continue de diviser nos deux chambres après l'échec de la commission mixte paritaire à propos des délits de presse, l'examen de cette proposition de loi a surtout permis de constater que la question de la temporalité de la justice est loin de faire consensus. En la matière, les aspirations de nos concitoyens sont parfois contradictoires. Les délais de l'instruction et du jugement leur semblent rarement satisfaisants. Lorsque la justice va vite, des voix s'élèvent pour dénoncer son caractère expéditif ; et lorsqu'elle va plus lentement, d'autres, parfois les mêmes, accusent les juges d'indigence. Il ne s'agit pas d'un sujet nouveau. Dès les années 2000, la bonne administration de notre justice a été mise en cause devant la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, et la France a été condamnée à de nombreuses reprises pour la lenteur de ses procédures judiciaires. Depuis lors, la jurisprudence des « délais raisonnables » s'est largement imposée dans notre droit, à budget constant. N'est-il pas paradoxal, au regard des efforts demandés aux agents chargés de l'instruction pour réduire les délais de jugement dans l'intérêt du justiciable, de permettre à ce dernier de se manifester des années, voire des décennies après la survenance de faits dont il s'estime victime ? Mes chers collègues, pour la prescription comme pour les délais de jugement, une seule question se pose à nous à quel moment la justice doit-elle être rendue pour être utile ? Tzvetan Todorov, disparu la semaine dernière, écrivait Le devoir de mémoire ne sera pas moralement justifié si le rappel du passé nourrit avant tout mon désir de vengeance ou de revanche, s'il me permet simplement d'acquérir des privilèges ou de justifier mon inaction dans le présent. Cette maxime pourrait également s'appliquer au requérant très tardif. En dehors des cas très particuliers que les juges prennent déjà en compte, à savoir les délits occultes et les omissions traumatiques, nous ne sommes pas favorables à une extension si longue du délai de prescription. Rappelons qu'il s'agit de doubler les délais de droit commun. Mes collègues Jacques Mézard et Jean-Claude Requier ont déjà évoqué les limites de cette initiative, également reconnues par nombre de magistrats, à commencer par les membres de l'Union syndicale de la magistrature et du Syndicat de la magistrature le dépérissement des preuves et la rancoeur contre le système judiciaire qui pourrait en résulter. Pour les éviter, il faudra peut-être songer à former nos juges aux techniques de l'archéologie Plus sérieusement, et alors qu'il s'agit probablement du dernier texte relatif à la justice pénale que nous examinerons sous ce quinquennat, nous regrettons que ce débat ne se soit pas inscrit dans une discussion plus large quant à la modernisation du code de procédure pénale et même de notre justice. Monsieur le garde des sceaux, vous n'êtes pas responsable de cette situation : vous avez pris le train des réformes en marche. Mais vous savez bien que ce débat s'impose depuis l'affaire d'Outreau et l'échec de la réforme de la collégialité de l'instruction. cours de ce quinquennat, un certain nombre de chantiers ont été ouverts afin de moderniser notre système pénal. La loi relative à l'individualisation des peines nous a permis de débattre de l'avenir des mesures alternatives aux peines de prison, qu'on les plébiscite ou que l'on s'y oppose. La nécessité de garantir l'indépendance de nos magistrats a également animé nos discussions, bien que certaines entreprises décrétales postérieures risquent de mettre à mal les maigres avancées obtenues en la matière. Nous avons tous à l'esprit les raisons qui, en revanche, nous ont contraints d'escamoter le débat sur l'amélioration de la procédure pénale : la nécessité de renforcer notre cadre légal de lutte contre le terrorisme. À nos yeux, les échanges que nous avons eus à ce sujet, en marge de l'examen de la loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, sont très insuffisants. Espérons que le prochain gouvernement se saisira de ce dossier Mes chers collègues, chacun de nous sait également que cette réflexion ne pourra déboucher sur des résultats probants si l'on maintient le ministère de la justice dans le carcan budgétaire qui est le sien. Là plus qu'ailleurs, on éprouve les limites de la théorie selon laquelle il est possible de faire mieux avec moins de moyens.

pour rendre notre système pénal plus efficace dans la lutte contre la récidive et plus respectueux des critères fixés dans nos engagements internationaux. Sans aller jusqu'aux solutions qui ont permis aux Pays-Bas de réduire drastiquement le nombre de leurs détenus, au point de louer une partie de leur parc carcéral à leurs voisins, notre réflexion pourrait se nourrir davantage des expériences étrangères. Enfin, l'examen de cette proposition de loi a mis en lumière le nouveau défi que nous pose internet, alors que certaines pratiques ravivent les débats relatifs à la liberté d'expression. Si, dans leur majorité, les membres du groupe du RDSE sont plutôt favorables à la rédaction proposée par le Sénat sur la question précise de la prescription des délits de presse sur internet, nous considérons que le sujet mériterait d'être approfondi dans un cadre plus large. Quoi qu'il en soit, cette préférence n'est pas de nature à emporter notre faveur pour l'adoption d'un texte dont- je l'ai dit -nous contestons le principe. La grande majorité des membres du groupe auquel j'appartiens voteront donc contre cette proposition de loi.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, nous voici réunis pour la troisième fois afin d'examiner la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale, après l'échec de la commission mixte paritaire réunie le 13 février dernier.

aux dispositions établissant l'imprescriptibilité de l'action publique pour les crimes de guerre connexes à un crime contre l'humanité. En effet, selon nous, le droit à l'oubli est un outil fondamental qui concourt à la pacification de notre société. De plus, nous avons fait valoir que ces dispositions risqueraient de banaliser le crime de génocide et les crimes contre l'humanité en rompant le caractère absolument exceptionnel de l'imprescriptibilité.

la proposition d'inscrire les plaintes simples parmi les actes interruptifs de la prescription, mesure contraire aux solutions retenues jusqu'à présent par la jurisprudence. Nous nous félicitons de toutes ces améliorations apportées à un texte que nous jugeons tout à fait important. Mais, malgré le large consensus qui s'est dégagé entre les parlementaires, nous nous sommes revus le 7 février dernier, parce que l'adoption définitive de cette proposition de loi avait achoppé en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, toutes les dispositions du présent texte bénéficient d'un accord entre les deux assemblées à l'exception d'une seule : celle qui est relative à la prescription des infractions de presse prévues par la loi de 1881, qui est aujourd'hui de trois mois.

et de l'action civile des abus de la liberté d'expression commis sur internet de trois mois à un an. Au nom de la défense de la liberté de la presse, les membres du groupe socialiste et les représentants du secteur de la presse en ligne se sont opposés à cette extension du délai de prescription du délit de presse. Pourtant, cette disposition s'expliquait, me semble-t-il, par le constat dressé par MM. François Pillet et Thani Mohamed Soilihi dans leur rapport d'information intitulé « L'Équilibre de la loi du 29 juillet 1881 1881 sur la liberté de la presse à l'épreuve d'internet » : l'insuffisante protection des victimes des abus de la liberté d'expression commis sur ce nouveau média.

à l'influence parfois plus grande sur le même réseau plusieurs mois plus tard, sans que la jurisprudence puisse considérer ces infractions de manière distincte. Dès lors, une personne peut aujourd'hui être victime de diffamations, d'injures ou de provocation à la haine ou à la discrimination qui, tout en étant en étant contemporaines, sont prescrites, puisque les messages litigieux ont été publiés pour la première fois plus de trois mois auparavant. Il y a là un véritable problème. L'excellent rapport de notre collègue François-Noël Buffet est venu à l'appui de cette position. En deuxième lecture, à l'Assemblée nationale, les députés Patrick Bloche et Isabelle Attard ont déposé un amendement visant à supprimer la disposition en question. Selon eux, cette mesure créerait une rupture d'égalité injustifiée dans le traitement réservé aux contenus diffusés sur supports papier d'une part, numérique d'autre part. Cet amendement a été adopté, le rapporteur Alain Tourret ayant estimé qu'il ne fallait pas modifier la loi de 1881 dans le cadre du présent texte.

décidé de rétablir le texte issu de ses délibérations au stade précédent de la navette, sous réserve de deux mesures de coordination. Ainsi, l'article 3 maintient à trois ans le délai de prescription de l'action de l'administration des douanes en matière contraventionnelle. Dans le même temps, il supprime la disposition, introduite par le Sénat, qui établit une différence de régime entre les infractions de presse qui sont commises sur support papier et celles qui sont commises en ligne. Sur ce point, la commission a retenu la version adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

le Sénat est saisi, en nouvelle lecture, de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale, après l'échec de la commission mixte paritaire réunie le lundi 13 février 2017. Ce texte, qui fait suite aux travaux conduits en 2015 par nos collègues députés Alain Tourret et Georges Fenech dans le cadre de la mission d'information sur la prescription en matière pénale, fait l'objet, sur un certain nombre de points, d'un large consensus entre les deux chambres Ainsi, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté dans des termes identiques les articles 1, 2, 4 et 5, qui ont vocation à moderniser le droit de la prescription.

Sur cette question particulière, que j'ai eu l'occasion d'aborder lors des précédentes lectures, le groupe écologiste n'est pas tout à fait convaincu. Bien sûr, le texte qui nous est soumis aujourd'hui a le grand mérite de poser le débat en termes généraux et de nous éloigner ainsi d'un droit d'exception que nous avons toujours refusé. Il renforce également la sécurité juridique en précisant clairement le point de départ du délai de prescription pour chaque infraction ou catégorie d'infraction. Mais si la nécessité de mettre à plat le droit de la prescription ne fait, pour nous, aucun doute, la nécessité d'allonger les délais de prescription de droit commun en matière délictuelle et criminelle ne nous semble pas aller de soi. Le Syndicat de la magistrature l'a rappelé hier dans une lettre ouverte adressée aux parlementaires : « les bonnes intentions ne feront pas une bonne législation ». Il affirme également, et nous partageons ces propos, que « la prescription n'est pas l'ennemie de la justice, elle est au contraire un de ses piliers. Garantie essentielle pour le procès équitable et surtout, condition de l'apaisement social que la justice recherche, elle procède d'un équilibre complexe. Malheureusement, ces considérations, pourtant capitales, ne sont plus l'objet de nos débats et nous ne discuterons aujourd'hui que de l'article 3, seul point de désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Cet article, rappelons-le, vise à faire passer le délai de prescription des infractions commises sur internet de trois mois à un an. La situation devient presque grotesque, mes chers collègues, puisque nous débattons de cette disposition exactement dans les mêmes termes que la semaine dernière. Je ne m'étendrai donc pas inutilement sur ce sujet, le groupe écologiste n'ayant pas changé d'avis depuis la dernière séance. Nous considérons que l'article 3, qui revient à créer deux délais de prescription pour une même infraction sur la base du support utilisé- internet seul ou internet et papier -, entache la lisibilité et la cohérence de la loi. Nous rejoignons ici la position de l'Assemblée nationale qui s'est prononcée hier et se prononcera à nouveau demain pour, probablement, défaire ce qui aura été fait aujourd'hui au Sénat.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme plusieurs orateurs l'ont dit avant moi, ce texte est très important pour le droit des victimes.

et il démontre que l'initiative parlementaire peut être très bénéfique- même s'il existe, monsieur le ministre, de bons ministres, qui préparent de beaux projets de loi

qu'il est possible, sur certains sujets, de dépasser les clivages habituels pour trouver d'utiles points de convergence.

un an, le maintien à trente ans du délai de prescription des crimes de guerre connexes à un crime contre l'humanité ainsi que- c'est important ! -le maintien du report du point de départ à la majorité pour les mineurs victimes de crimes et délits

J'en viens maintenant au seul point de désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, même si, monsieur le président Philippe Bas, je tiens à saluer ceux qui se sont employés à trouver un compromis, sans y parvenir.

Jacques Bigot, Alain Richard et René Vandierendonck partagent, sur la question des délits de presse et des délits sur internet, la position de la majorité du Sénat et de la commission des lois. Notre groupe, dans sa grande majorité, c'est-à-dire tous ses autres membres, a choisi, après réflexion, de soutenir la position de l'Assemblée nationale et du Gouvernement, pour des raisons assez simples et que je vais redire ici. Sur le plan juridique, vous le savez, le principe de la neutralité de support prévaut depuis très longtemps pour la réglementation et la régulation dans l'ensemble du secteur des communications audiovisuelles, télécoms et nouveaux médias.

Au titre de cette neutralité technologique, la fiscalité de la presse en ligne a d'ailleurs été alignée sur celle de la presse papier, au taux de 2,1 %. La loi sur la presse a déjà été modifiée afin d'allonger la prescription pour certaines infractions, mais sans faire de différence entre les supports. supports. La distinction effectuée par la majorité de la commission des lois et du Sénat lui-même entre le régime applicable, d'une part, à la presse sur papier et et à la presse en ligne reproduisant des articles publiés dans la presse papier et, d'autre part, à la presse en ligne ne prend pas véritablement en compte l'évolution de la profession journalistique. Les journalistes, que nous avons bien sûr disent que la réalité actuelle de leur travail et des rédactions conduit à publier indifféremment, toutes les heures du jour et de la nuit, sur des supports papier et sur des supports numériques, sans qu'un auteur sache, au départ,

ouvrage, reproduit sans qu'il soit question de rémunérer l'auteur, celui qui a travaillé. Hélas ! Les mêmes débats ont lieu dans le domaine artistique et dans le domaine de la culture.

c'est l'anonymat sur internet. Aujourd'hui, il existe des milliers, voire des dizaines ou des centaines de milliers de messages qui n'ont pas d'auteur.

justice ! -d'évoquer la position d'une minorité de nos collègues et la position de la majorité de nos collègues, notre groupe votera l'amendement que va présenter dans un instant Mme Esther

J'ai eu l'occasion de le dire lors de la discussion générale, le groupe écologiste considère que rien ne justifie l'allongement de trois mois à un an du délai de prescription des infractions commises par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. Dans un texte qui vise d'abord à rendre le droit de la prescription plus cohérent et plus lisible, la création de deux délais de prescription pour une même infraction en fonction du support utilisé nous semble tout à fait contre-productive. Nous considérons également, à l'instar du Gouvernement, que toute modification de la loi de 1881 doit être envisagée avec une très grande Il ne s'agit de rien de moins que du fragile équilibre entre liberté d'expression et répression des abus de cette liberté. Si une réforme de cette loi s'avère nécessaire à l'heure du numérique, il convient d'y apporter rigueur et réflexion approfondie.

de la commission ? La commission s'est prononcée plusieurs fois sur cet amendement au fil de la procédure, à chaque fois négativement. Je ne puis donc que réitérer cet avis défavorable, pour les motifs que j'ai exposés dans la discussion générale.